rappel au règlement

La Russie et l'Ukraine sont en guerre depuis plus d'un an et, plus inquiétant encore, plus ça va, plus la France s'engage et devient un cobelligérant, comme d'ailleurs les autres pays de l'Union européenne.

sur ce sujet. En effet, on ne peut pas laisser le Gouvernement faire ce qu'il veut, au prétexte que c'est lui qui, de par la Constitution, décide. C'est vrai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

Je rappelle par exemple que nous devons la création de la Caisse des Français de l'étranger à notre ancien collègue Jean-Pierre Cantegrit. Plus récemment, la proposition de loi de Bruno Retailleau, votée il y a bientôt trois a balayé de nombreux sujets au coeur des préoccupations des Français établis hors de France, notamment un volet sur la fiscalité de leur résidence en France. Permettez-moi également d'évoquer notre proposition de loi, votée à l'unanimité le 30 juin 2020, portant création d'un fonds d'urgence pour les Français de l'étranger victimes de catastrophes naturelles ou d'événements politiques majeurs.

Enfin, je tiens à remercier l'ensemble des membres de la commission des finances et son président, qui ont adopté mercredi dernier en commission le texte que nous débattons aujourd'hui.

Par un hasard étonnant, qui n'a certainement rien à voir avec le fait que notre proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour des travaux du Sénat, le Gouvernement annonce la semaine dernière la mise en place de ce groupe de travail qu'il en soit, retenons ceci : nous, sénateurs, faisons bouger les choses ! Nous obligeons le Gouvernement à répondre aux avancées que le Sénat propose. Seule la défense de l'intérêt général guide nos travaux. La proposition de loi que nous étudions aujourd'hui répond à une demande récurrente et ancienne des Français de l'étranger, au-delà des considérations partisanes. Il existe plusieurs catégories de Français établis hors de France. Il y a ceux qui sont nés à l'étranger, pour la deuxième, parfois la troisième génération. Il y a ceux qui quittent la France pour tenter leur chance, créer une entreprise, enseigner, être salariés, faire rayonner la culture française à l'étranger. Il y a ceux qui rencontrent un conjoint étranger et le suivent dans son pays. Il y a ceux qui choisissent de vivre une partie de leur retraite à l'étranger. Il y a aussi ceux, nombreux, qui s'expatrient quelques années par obligation professionnelle. Partout, quelles que soient les situations- et elles sont multiples -, les Français qui vivent à l'étranger font rayonner la France dans le monde. Pensez un instant à cet entrepreneur français qui importe des produits fabriqués en France pour les vendre dans son pays de résidence. Non seulement il profite au commerce extérieur, mais, bien au-delà, il crée des emplois sur le territoire national ! Les professeurs français qui enseignent le français à l'étranger font rayonner notre langue et notre culture.

établis hors de France gardent des liens forts avec la France, leur patrie, leur famille, leurs amis. Nombre d'entre eux y reviennent régulièrement. Nombre d'entre eux y ont une maison de famille, qui est leur port d'attache et qu'ils souhaitent conserver, parfois pour y revenir finir leur vie et la transmettre à leurs enfants. Et que dire de ceux qui vivent dans des zones dangereuses ou qui se retrouvent pris dans une guerre ? Mes collègues sénateurs représentant les Français établis hors de France et moi-même avons eu à gérer des situations de retour en urgence en France de compatriotes pris dans la tourmente.

argument ! Pensez aux Français du Burkina Faso, qu'ils vivent à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso. Vous savez que les autorités de ce pays ont demandé que les troupes françaises quittent

Aujourd'hui, nombre de nos compatriotes qui vivent à l'étranger et qui sont dans ces situations doivent se séparer de leur résidence en France, parce que la fiscalité est trop lourde pour eux. Il s'agit souvent d'une maison familiale

La France doit permettre aux Français de l'étranger de garder une résidence en France. Elle doit aussi inciter ceux qui n'en ont pas encore d'en acquérir une, ce qui ferait revenir des capitaux français dans notre pays.

nous obligeons le Gouvernement à aller jusqu'au bout. Nous posons le principe de la création du statut de résidence d'attache- ce terme montre combien il est question d'attachement à la France. Par l'amendement que je présenterai tout à l'heure, nous ne permettrons pas au Gouvernement d'enterrer les conclusions du groupe de travail. Aujourd'hui, le Sénat a une nouvelle fois l'occasion de démontrer qu'il est bien la « maison des Français de l'étranger ». Nous répondrons à une demande forte de ces Français et nous répondrons aussi à l'intérêt de la France.

2,5 millions de Français hors de France : ce ne sont pas des sous-Français, ce sont des Français à part entière. Comme Ronan Le Gleut vient de le souligner, ils participent à la grandeur de la France, comme nos outre-mer, que nous oublions trop souvent dans nos textes. Au Sénat, nous n'oublions personne. Ces 2,5 millions de Français sont au coeur de nos préoccupations. Cela fait plusieurs années que, sur toutes les travées, en particulier sur celles

secondaire. Les Français de l'étranger ne sont pas toujours ce que l'on appelle des expatriés, c'est-à-dire ces Français parfois un peu privilégiés envoyés par de grandes entreprises ou par l'État, l'État, moyennant des conditions financières plutôt avantageuses et un déroulement de carrière favorable. Ce sont parfois aussi des Français qui sont obligés de quitter leur pays pour des raisons diverses et variées, ne serait-ce que parce que leur conjoint est

En suivant l'actualité de l'Assemblée nationale, nous avons compris qu'un député de la majorité- relative - du Président de la République, Frédéric Petit, s'intéressait également

les résidences secondaires (THRS). Nous nous sommes adaptés à la suppression de la taxe d'habitation, décidée par le Président de la République, que les maires de France regrettent- non pas le Président de la République, mais la taxe d'habitation.

dans ce texte sont bienvenues : créer le statut de résidence d'attache pour répondre à une demande ancienne et légitime et créer un statut qui pourrait à l'avenir servir de support de politiques publiques en faveur des Français de l'étranger. Voilà ce qui nous manque.

entre nos deux pays, j'ai réuni les communautés françaises de New York et de Washington : c'est toujours une très grande fierté pour un ministre de la République que de rencontrer ces Français qui font rayonner notre pays bien au-delà de nos frontières. Avant d'aborder le coeur du dispositif proposé par Ronan Le Gleut, ainsi que les modifications apportées par le rapporteur Jérôme Bascher, permettez-moi de rappeler des points essentiels. essentiels. Je le dis sans ambages : nous sommes fiers de celles et ceux qui réussissent ailleurs et nous devons les y aider. Nous devons être à leurs côtés, parce que, quand ils réussissent, c'est aussi la France qui réussit.

Je pense par exemple aux questions de simplification des démarches administratives. À ce titre, je rappelle un certain nombre de mesures très concrètes

taxe -, la dématérialisation de la délivrance d'extraits et de copies d'actes ou, bien sûr, la création de la plateforme France Consulaire, en cours de déploiement. Je pense aussi au soutien massif apporté à nos compatriotes qui étaient à l'étranger pendant la crise covid. Ce sont ainsi 220 millions d'euros qui ont été mis sur la table en urgence pour les aider à surmonter ce moment incroyablement difficile, mais aussi pour mettre en place des services de téléconsultation ou des aides au rapatriement. Les sujets de fiscalité ne sont pas en reste, puisque nous avons aussi permis d'importantes avancées au cours des dernières années, notamment au travers de la loi de finances pour 2021. Ce texte a, par exemple, prévu la déduction, sous certaines conditions, des pensions alimentaires versées par les contribuables non-résidents non-résidents ou l'exonération de plus-values immobilières pour les contribuables qui transfèrent leur résidence fiscale hors de France, si la cession intervient au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit le départ. Pour autant, je suis conscient qu'il nous reste du chemin à parcourir en matière de simplification fiscale pour les non-résidents. Le renforcement très significatif des moyens de la DINR, intervenu durant

les tentatives que nous avons conduites pour introduire davantage d'automaticité dans le prélèvement de l'impôt pour les non-résidents se sont heurtées à la complexité inhérente à l'application de multiples conventions fiscales.

d'un engagement du Président de la République. Celui-ci s'est déclaré favorable à l'inscription dans notre droit de la notion de « résidence de repli »- ou de « résidence d'attache » pour reprendre les termes de la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui. Quel est le cadre actuel ? Depuis cette année, plus aucune résidence principale n'est assujettie à la taxe d'habitation, ce qui est une bonne nouvelle pour les contribuables français. Celle-ci reste toutefois due au titre des résidences secondaires et, plus généralement, des locaux meublés destinés à un usage autre que d'habitation principale. Ainsi, les locaux d'habitation situés en France et détenus ou loués par des Français résidant ordinairement dans un autre logement, en France ou à l'étranger, sont regardés comme des résidences secondaires, dans la mesure où ils ne répondent pas aux critères retenus par l'administration fiscale pour qualifier un logement de résidence principale. Les résidences secondaires Les résidences secondaires sont également susceptibles de se voir appliquer la majoration de taxe d'habitation prévue en zone urbaine tendue ou, en application de la loi de finances pour 2023, dans les communes touristiques présentant des critères de tension immobilière. Cette majoration est fixée par les communes à un taux variant de 5 % à 60 %. Elle a pour finalité d'inciter à ce que des logements sous-occupés soient remis sur le marché, uniquement dans les zones où de fortes tensions sur le marché du logement le justifient. Pour rappel, on estime à près de 300 000 le nombre de résidences secondaires dont le propriétaire réside hors de France, sans que l'on soit en mesure de savoir si

liée auxdites résidences représente un montant total de 340 millions d'euros d'impôts locaux. Le texte qui nous occupe a été profondément remanié par M. le rapporteur Jérôme Bascher, dont je souhaite saluer l'ampleur du travail.

D'une part, le statut de résidence d'attache entraînerait l'exemption de majoration de la THRS dans les zones tendues. D'autre part, le texte prévoit l'application d'un dégrèvement

Pour autant, le statut fiscal de la résidence de repli soulève des questions juridiques majeures éminemment complexes et un risque élevé de non-conformité au droit européen et à la Constitution.

En particulier, au lieu d'aider à la prise en charge des frais de rapatriement lorsqu'ils excèdent les capacités financières du contribuable, l'avantage fiscal dépendrait, d'une part, du taux appliqué par la commune et, d'autre part, de la valeur du bien. Son montant serait donc sans lien avec le risque auquel est exposé le Français de l'étranger bénéficiaire de l'avantage fiscal ni avec les coûts liés à son retour en France.

a vocation à aborder le sujet de la résidence d'attache sous l'angle fiscal, mais aussi non fiscal, ainsi que toute autre mesure susceptible de soutenir les Français de l'étranger face aux risques auxquels ils sont exposés.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, tous les Français ont un coin de France qui leur est cher. C'est souvent le lieu de leur enfance, toujours un endroit où ils nouent attache avec leur pays. C'est généralement dans ce lieu que nos compatriotes souhaitent posséder une résidence. Elle matérialise ce puissant lien d'affection avec le pays. Cet appartement ou cette maison ne se situe pas toujours dans une grande ville ou dans une zone tendue. Il s'agit parfois d'un bien familial, situé dans un petit village au coeur de nos campagnes. Cette résidence a une valeur spéciale pour chaque Français. Cela vaut tout particulièrement pour nos compatriotes expatriés. Pour eux, cette résidence est un ancrage avec le territoire, une attache avec le pays. Lorsqu'ils reviennent en France, par choix ou par contrainte, cette résidence est pour eux un point de retour. C'est pourquoi notre groupe accueille avec bienveillance l'intention de cette proposition de loi, qui vise à reconnaître le statut particulier de cette résidence. n'est ni une résidence principale, puisque ces Français n'y ont pas établi leur domicile, ni tout à fait une résidence secondaire, puisqu'elle peut être amenée à redevenir une résidence principale dès que l'expatriation prend fin. Sur ce point, les cas de figure soulevés par les auteurs du texte ne peuvent laisser insensibles. Je pense notamment à nos compatriotes qui vivaient en Ukraine au moment où la Russie a lancé son offensive absurde et sanguinaire, et qui ont dû être rapatriés en urgence pour fuir l'horreur de la guerre. Pour eux, la maison ou l'appartement qu'ils possèdent en France est effectivement devenu un refuge. Que ces Français soient traités par les services fiscaux comme des citadins en escapade, pour une partie de campagne ou un week-end à la mer, a en effet de quoi surprendre. C'est pourquoi cette proposition de loi nous invite à créer une nouvelle catégorie de résidence fiscale, permettant un traitement différencié. L'article 1, qui crée cette nouvelle catégorie de résidence, ne pose pas de difficultés. Il nous est proposé d'appeler cette résidence « résidence d'attache », ce qui est assez élégant. Le Président de la République, qui avait fait une promesse de campagne voisine, avait opté pour « résidence de repli », ce qui est plus précis. Quelle que soit l'épithète retenue, notre groupe n'est pas hostile à la création de cette catégorie, qui correspond à une demande formulée depuis plusieurs années par les expatriés. Elle a certes l'inconvénient d'ajouter un nouvel article au code général des impôts et donc de la complexité à notre droit. Or c'est par la superposition des bonnes intentions que l'on crée des monstres juridiques tels que nos codes de droit.

Sur ce point, on ne peut se contenter, pour légiférer, de s'intéresser aux cas extrêmes, comme celui des Français en Ukraine, confrontés à l'horreur de la guerre. Nous devons aussi considérer le cas de tous les expatriés qui ont fait le choix de l'expatriation, le plus souvent pour leur carrière. Ceux-là obtiennent généralement, par les conditions de leur expatriation, des compensations à la hauteur des contraintes auxquelles ils consentent en vivant loin de la France.

C'est pourquoi je me réjouis que la commission des finances ait joué son rôle de gardienne des deniers publics, en limitant l'impact financier de ce texte. En remplaçant le mécanisme d'exonération par un dégrèvement et en limitant l'éligibilité aux seuls expatriés contraints de revenir en France à cause de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté, le dispositif se concentre désormais sur les cas de figure qui ne font pas débat.

que vous avez présentés pour nous proposer de réfléchir plus longuement aux conditions posées par ce texte. Néanmoins, pour toutes les raisons que j'ai exposées et sous réserve d'une réflexion future, notre groupe ne peut être hostile à à cette proposition de loi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Augustin est brutalement réveillé par de violentes secousses. Un mur de sa chambre s'effondre, le plafond s'ouvre. Dans ce double tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie, plus de 53 000 personnes ont trouvé la mort, dont 8 Français. Augustin est chanceux, il sort vivant de cette catastrophe.

locative. Le besoin d'aider au retour des Françaises et Français qui souhaitent rentrer en France existe donc bel et bien, en particulier lorsqu'ils et elles vivent dans des pays en crise et que ce besoin de retour est, par définition, soudain et urgent.

mesure où seuls les logements non loués pourraient être déclarés comme résidence d'attache, une telle catégorie bénéficierait aux personnes qui font le choix de laisser leur logement vide, ce qui n'est évidemment pas le sens des politiques de logement que nous devons mener.

supprimer les discriminations fiscales à l'encontre des Français de l'étranger, par exemple pour les rénovations ou pour les dons aux associations. En

rattacher l'une de leurs résidences à ce statut. Elle tend également à leur accorder une exonération de taxe d'habitation. Le Président de la République s'était engagé, lors de la campagne présidentielle, à créer une notion de « résidence de repli » à laquelle s'attacheraient « certains avantages de la résidence principale La création de cette notion répond notamment au besoin de protection et d'accompagnement des Français établis hors de France, qui peuvent être menacés par des crises de nature sanitaire ou encore géopolitique, comme l'irruption d'un conflit armé sur le sol européen nous l'a récemment rappelé.

de pouvoir revenir en urgence si des circonstances exceptionnelles le justifiaient. Ainsi, l'article 1 institue la catégorie de résidence d'attache et prévoit les modalités par lesquelles les Français établis hors de France qui possèdent ou louent un logement secondaire en France peuvent- pour l'un de leurs biens seulement -revendiquer ce statut. Nous pouvons cependant nous étonner qu'aucune des conditions ni aucun des droits attachés à ce nouveau statut ne soient définis dans cet article et que ses modalités et conditions d'application soient renvoyées à un simple décret. En outre, un tel dispositif risque, s'il est insuffisamment encadré, de causer une rupture d'égalité avec des résidences secondaires qui répondraient aux mêmes caractéristiques que la résidence d'attache. Il risque également d'être contraire au droit européen, en privilégiant certains contribuables non-résidents, en raison de leur nationalité.

THRS valable un an, pour la résidence de repli des Français contraints au rapatriement « en raison de la survenue d'un événement extérieur à leur volonté dans leur pays d'accueil qui met en danger leur vie ou celle de leur famille ou qui y rend matériellement impossible une habitation durable ». Cette solution, bien qu'elle permette d'encadrer le dispositif, présente deux défauts majeurs. la majoration de THRS applicable en zone tendue est défendue par les élus locaux comme un outil d'aménagement et de revitalisation du territoire communal. Dans les zones où la part de résidences secondaires pèse sur le dynamisme de la commune, il permet d'inciter les propriétaires à habiter les logements ou à les mettre en location.

concerne la THRS et s'applique à la résidence de repli des Français contraints au rapatriement. Or, en cas de rapatriement, il est nécessaire de régulariser sans délai sa situation fiscale, ce qui implique de déclarer une nouvelle résidence principale qui remplacera ainsi la résidence de repli. Cette disposition est donc inopérante. Enfin, cette proposition sélectionne grandement les Français établis hors de France concernés par la mesure. En effet, les conditions à réunir pour déclarer cette résidence d'attache- posséder un bien en France qui ne génère pas de revenus locatifs -ne permettent pas de cibler tous les Français établis hors de France.

est forte, mais manifestement contraire à notre Constitution et aux engagements de la France. Chaque fois, la solution qui nous est proposée est une réécriture, qui, au bout du compte, ne peut satisfaire personne. Mes chers collègues, il est essentiel

et nous nous rallierons au travail qui vient d'être lancé par le Gouvernement sur ce sujet. Il associera les élus, dont les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, avec la ferme intention d'aboutir. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons cet après-midi une proposition de loi qui vise à compléter le droit des statuts fiscaux en créant un nouveau statut, celui de résidence d'attache.

Si le bien produisait des revenus locatifs, la taxe applicable aux locataires serait de fait la taxe d'habitation sur les résidences principales, aujourd'hui supprimée. Les biens mis en location

la généralisation de cette mesure serait inéquitable et probablement inconstitutionnelle. Elle viendrait rompre l'égalité de traitement au détriment de nos concitoyens vivant en France et possédant une résidence secondaire. Elle encouragerait par ailleurs le maintien de nombreux logements vides, alors que l'on connaît l'ampleur de la crise du logement dans notre pays et que nous devons tout faire pour la résoudre. Elle créerait aussi un lien très général, et peut-être dangereux dans ses conséquences, entre nationalité et fiscalité. elle pourrait peser lourdement sur les finances publiques, sans aucune nécessité puisque l'immense majorité de nos compatriotes établis à l'étranger vivent dans des pays où leur sécurité n'est pas menacée.

vous le dites vous-même dans l'exposé des motifs, cher Ronan Le Gleut, les conflits en Ukraine et dans la région du Tigré sont de récents exemples de la nécessité de prévoir une résidence d'attache, de refuge ou de repli. On peut penser aussi à un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, où la situation est particulièrement instable. C'est pourquoi, pour nous prononcer favorablement sur ce texte, nous souhaitons ajouter comme condition préalable au dégrèvement de THRS le fait de résider dans un pays classé par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères Cela réserverait le bénéfice de cet avantage fiscal à nos concitoyens vivant dans des pays très risqués et vaudrait pour la THRS comme pour l'exonération totale en cas de retour précipité et contraint.

Pour résumer : oui à une résidence d'attache, bénéficiant d'un avantage fiscal, pour nos compatriotes vivant à Kiev ou à Ouagadougou, mais seulement pour eux, car ils sont les seuls à avoir besoin d'un refuge, qu'ils le mobilisent ou non dans l'année fiscale. Voilà notre réaction à ce texte : vigilante, mais aussi très constructive. J'espère que nos travaux nous permettront, en délimitant précisément la notion de résidence d'attache comme un véritable refuge,

les Français ayant choisi de s'expatrier doivent avoir le moins possible de relations fiscales avec la Nation. Autrement dit, toute contribution qui leur serait demandée mériterait d'être diminuée, voire supprimée. On est très loin de l'aide au retour ...

se situent trop souvent dans des zones tendues, où le manque d'habitations est important et où le prix de l'immobilier explose. Mais les règles fiscales devraient, selon vous, être différentes selon qu'on est d'un côté ou de l'autre de la frontière.

Votre objectif, selon l'exposé des motifs, est que « cette résidence constitue un point d'attache avec la France, qui les relie à leur famille et à leur patrie ». Dès 1983, le Conseil constitutionnel a fondé son contrôle sur les « critères objectifs et rationnels » de la différence de traitement sur le plan fiscal.

concrets : il s'agit de quelques centaines d'euros par année, alors que d'autres types d'hébergement- résidence chez la famille ou les amis, hôtel, location, accueil solidaire -permettent aux Françaises et aux Français expatriés de s'établir temporairement en France, pour ceux qui n'auraient pas les moyens de s'acquitter d'une telle taxe. taxe. Au risque de vous choquer, dois-je vous rappeler qu'à l'heure où vous vous préoccupez de ceux qui sont propriétaires, mais ne résident pas dans leur logement, seuls 38 % des résidents en France sont propriétaires non-accédants, c'est-à-dire sans crédit à supporter. Pis, 14 % des résidents en France disposeraient d'un autre logement en France, 4,9 % d'une résidence secondaire. Votre proposition n'est finalement ni plus ni moins qu'un moyen de consacrer les inégalités. ne serait que regrettable si ce n'était habituel. Alors que la concentration du patrimoine immobilier s'est accrue depuis 2000 de 125 milliards d'euros, dont la moitié résulte de l'augmentation de la part détenue par les non-résidents,

contre 69 998 euros pour les résidents. Mes chers collègues, cette proposition de loi créerait un effet d'aubaine pour les plus fortunés, ceux qui connaissent le mieux la fiscalité- car votre déclaration, si j'ai bien compris, se ferait sur demande.

Ces résidences sont actuellement considérées par le droit fiscal comme des résidences secondaires, et sont par conséquent assujetties à la taxe d'habitation. Il est vrai que les propriétaires de résidences secondaires sont particulièrement exposés à la fiscalité locale,

Nous l'avons dit et redit, mais c'est l'occasion de le répéter : la suppression de la taxe d'habitation sur la totalité des résidences principales non seulement a réduit l'autonomie fiscale des collectivités locales- une autonomie responsable, en ce sens que le choix du niveau de dépenses avait une conséquence directe sur les impôts des électeurs locaux -, mais elle a de surcroît relâché presque totalement le lien démocratique, en dissolvant le contrat local entre citoyens et élus, entre taxation et représentation, qui n'a apparemment pas de valeur constitutionnelle en France

-a proposé d'y substituer un dégrèvement pris en charge par l'État l'année du retour d'un Français de l'étranger, lorsque ce retour est justifié par la survenue d'un événement extérieur à la volonté de celui-ci, qui met en danger sa vie ou celle des membres de sa famille ou qui rend matériellement impossible son habitation dans le pays d'accueil.

Le resserrement du périmètre de l'allégement fiscal se justifie aussi pour des raisons constitutionnelles, qui imposent de respecter le principe d'égalité devant les charges publiques. Mais pourquoi n'accorder ces avantages fiscaux qu'aux seuls Français résidant à l'étranger ? « Privilège suppose quelqu'un pour en jouir et quelqu'un pour le payer », écrivait Frédéric Bastiat. Je suis, pour ma part, à l'image de ma collègue Vanina Paoli-Gagin, attaché au caractère universel de la loi, y compris la loi fiscale. Ces avantages catégoriels, ciblés- probablement un hasard -à quelques mois des élections sénatoriales, sur les seuls Français résidant à l'étranger, nous semblent nuire tout à la fois aux finances publiques, à l'égalité devant l'impôt et à la clarté du système fiscal. Par ailleurs, le ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, Olivier Becht, a indiqué il y a tout juste une semaine que les parlementaires représentant les Français de l'étranger, dont notre collègue Olivier Cadic, allaient examiner la proposition du Président de la République, Emmanuel Macron lui-même, qui, pendant la campagne présidentielle, s'était engagé à créer un statut de résidence de repli. L'objectif de ce groupe de travail, qui vous a été confié, monsieur le ministre, et auquel nous participerons, est d'arrêter dans un premier temps une définition de la notion de résidence d'attache, ou de repli. Ce n'est qu'une fois cette définition arrêtée que la résidence d'attache ou de repli devrait être assortie d'un régime fiscal adapté, vraisemblablement à l'occasion du projet de loi de finances pour 2024.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la décision de supprimer la taxe d'habitation a été une mesure à la fois aberrante, démagogique et profondément injuste. d'une part, parce qu'elle a privé les collectivités locales de ressources financières autonomes, d'autre part, et surtout, parce qu'elle fait dorénavant reposer la fiscalité locale sur des décisions prises par des gens qui ne la supportent pas,

Cette mesure était aussi profondément injuste. L'illustration de cette injustice est apportée par la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui. En effet, il n'y a pas de raison de faire une différence de traitement entre une résidence principale et la résidence de sauvegarde d'un Français qui réside à l'étranger, surtout lorsqu'il y a des

l'application parfois trop systématique et trop restrictive de l'article 45 de la Constitution, qui nous empêche d'examiner un certain nombre d'amendements.

ces mots qu'un lien charnel avec la mère patrie persiste chez de nombreux concitoyens installés à l'étranger ? Aujourd'hui, environ 1,7 million de personnes sont inscrites au registre des Français établis hors de France, mais les autorités estiment leur nombre total à près de 2,5 millions. Par comparaison, près de 3 millions de nos concitoyens vivent dans des départements et collectivités d'outre-mer. Les profils des expatriés sont divers, mais, parmi les personnes enregistrées, les adultes avec enfants et les seniors sont nettement majoritaires. La majorité d'entre eux sont installés à l'étranger pour des séjours de longue durée, et près de la moitié possèdent une autre nationalité. Pour beaucoup, l'expatriation apparaît donc comme un mode de vie à part entière. ils sont représentés par l'Assemblée des Français de l'étranger. Ils élisent également des représentants à l'Assemblée nationale depuis 2012, et depuis 1946 au Sénat- à l'époque Conseil de la République. Leur participation aux élections reste toutefois plus faible que la moyenne, pour des raisons à la fois politiques et pratiques. Par définition, les Français établis hors de France ne peuvent avoir leur résidence fiscale en France. Celle-ci n'a d'ailleurs pas de lien avec la nationalité : selon le code général des impôts, une personne est considérée comme résidant fiscalement en France si son foyer ou lieu de séjour principal est situé en France, si elle travaille en France, ou bien si le « centre de ses intérêts économiques se trouve en France ». Les agents publics exerçant à l'étranger sont considérés comme résidant en France s'ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dans leur pays de résidence. La réforme de la taxe d'habitation, lancée en 2018, s'est achevée cette année avec, depuis le 1 janvier, la suppression de l'imposition sur les résidences principales pour l'ensemble des ménages. La question de la compensation des pertes de recettes pour les communes et les intercommunalités a été maintes fois abordée, et l'on pouvait s'attendre à des répercussions de la réforme sur la taxe foncière et la THRS. Dans l'imaginaire collectif, la résidence secondaire Dans l'imaginaire collectif, la résidence secondaire est souvent associée à la maison de vacances, qu'il s'agisse d'une maison à la campagne, au bord de la mer, à la montagne ou d'un simple pied-à-terre dans une grande ville. Comme dans bien d'autres domaines, le fisc, lui, ne fait pas de sentiment, et il ne distingue pas, parmi ces résidences, celle qui peut aussi être la maison de famille. Lors de l'examen de la dernière loi de finances, il a été question de la nouvelle articulation à trouver entre la taxe foncière et la THRS, comme la taxe d'habitation sur la résidence principale a disparu en tant qu'impôt local de référence. Les amendements adoptés au Sénat n'avaient finalement pas été conservés en nouvelle lecture. N'oublions pas non plus la taxe sur les logements vacants, qui peut s'appliquer dans les zones résidentielles tendues. Dans ce contexte, la présente proposition de loi suscite quelques interrogations. La version initiale prévoyait une exonération pure et simple de la taxe d'habitation pour les Français non-résidents déclarant une résidence d'attache, catégorie nouvellement créée et dérogeant à la définition commune de la résidence fiscale. La semaine dernière, la commission des finances est allée dans la bonne direction en resserrant le dispositif : l'exonération est devenue une non-majoration de la taxe d'habitation, et un dégrèvement spécifique a été introduit pour leur année de retour au bénéfice des Français qui seraient contraints de revenir en France, notamment en cas en cas de perte d'emploi, de guerre ou d'autre catastrophe. Si ce dernier cas s'est produit récemment avec les conflits en Ukraine ou en Éthiopie, on peut se demander si le dispositif demeure parfaitement adapté à un tel objectif, en particulier la non-majoration. Par ailleurs, la question de sa pertinence vis-à-vis des autres catégories de contribuables, comme les résidents français ou bien les propriétaires étrangers, peut se poser. C'est pourquoi

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi créant une résidence d'attache pour les Français établis hors de France, portée par notre collègue Ronan Le Gleut, est une demande ancienne de la part des représentants- de tous bords politiques -des Français établis hors de France. « Sur le dossier fiscal fondamental de la résidence unique que certains possèdent en France et qui représente un lien solide avec notre pays, le groupe de travail " fiscalité ", mis en place en novembre 2004, a obtenu l'appellation " habitation unique en France ". Par souci d'égalité, nous agirons pour que vous soyez soumis à l'avenir aux mêmes impositions et aux mêmes taxes que les Français de métropole pour votre habitation en France. Demande récurrente également, donc, car les mots que je viens de prononcer sont ceux du candidat Nicolas Sarkozy dans sa lettre adressée aux Français de l'étranger le 30 mars 2007.

pour les Français de l'étranger victimes de catastrophes naturelles ou d'événements politiques majeurs », adoptée par le Sénat à l'unanimité, sur proposition de notre collègue Ronan Le Gleut le 30 juin 2020. Sous une forme juridique ou une autre, que son appellation soit « habitation unique », « résidence de repli », « résidence d'attache » ou « résidence de refuge », le sujet est abordé depuis de nombreuses années. Pour de sombres raisons, sur lesquelles je ne reviendrai pas, le statut fiscal de l'habitation unique a été dévoyé et s'est d'ailleurs assorti depuis 2012 d'une batterie de nouvelles taxes et impôts, dont les Français de l'étranger ont été les cibles. Inutile de vous rappeler l'épisode de la CSG-CRDS La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui permettrait à nos compatriotes expatriés de bénéficier d'un dégrèvement de la taxe d'habitation sur leur résidence située en France. Sous une forme ou une autre, cet aménagement a toujours été compris et adopté

J'y apporte bien évidemment tout mon soutien et celui du groupe Les Républicains, car, comme l'a très justement rappelé notre collègue Ronan Le Gleut, la résidence en France de nos compatriotes de l'étranger n'est pas qu'un lieu de villégiature pour exilés fiscaux ; c'est un véritable port d'attache, qui n'a rien de secondaire, notamment en cas d'urgence. Sous certaines conditions, cette résidence de repli, voulue par le Président de la République, ou d'attache, appellation qui me semble plus pertinente et plus concrète, ne peut souffrir d'une rupture d'égalité au regard, notamment, de l'assujettissement à la taxe d'habitation. Jusque-là, tout va bien. Même si je ne suis pas né de la dernière pluie, j'ai entendu les réticences de certains, fondées sur la crainte d'une possible inconstitutionnalité du texte. Je regrette néanmoins que la proposition de loi présentée aujourd'hui se retrouve quelque peu allégée, malgré le fait le fait que le Sénat en ait adopté à de nombreuses reprises le fond, comme le président Retailleau peut le confirmer. Je tiens à saluer ici le travail du rapporteur Jérôme Bascher, qui a su, malgré de nombreuses contraintes, proposer un dispositif qui n'est pas aussi ample, mais qui marque une avancée notable en faveur de nos compatriotes de retour en France qui, « en raison de la survenue d'un événement extérieur à leur volonté dans leur pays d'accueil qui met en danger leur vie ou celle de leur famille ou qui y rend matériellement impossible une habitation durable, ont été ont été contraints de venir résider dans leur résidence d'attache ». Il n'en demeure pas moins que des interrogations subsistent, et elles sont légitimes. Pourquoi une résidence non louée, seul lien avec la France- et, encore une fois, port d'attache de nos compatriotes -n'entrerait-elle pas dans le dispositif que propose la commission ? Concomitamment, signe de la pression exercée par le Sénat sur le Gouvernement depuis que nous avons lancé l'alerte sur la question de la résidence d'attache, la mise en place d'un groupe de travail sur cette question est désormais acquise et placée sous votre tutelle, monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics. Ce texte représente une avancée, ne nous le cachons pas, mais une avancée plus modeste que nous ne l'aurions souhaité, ne nous le cachons pas non plus. C'est dire, monsieur le ministre, que le groupe de travail- le énième qui est mis en place depuis quinze ans que je suis élu

en négatif. Puis, notre pays doit respecter le droit européen. Qu'en serait-il des ressortissants de l'Union européenne qui auraient une résidence dans notre pays ? Faudrait-il les traiter comme des Français ?

cet objectif de solidarité avec les remarques qui ont pu être faites en matière d'égalité devant l'impôt et de droit européen. Nous saluons le travail du rapporteur sur ce point, même si nous considérons que celui-ci mérite d'être encore affiné. D'abord, un dégrèvement global nous semble

Beaucoup d'entre eux restent propriétaires d'une résidence en France. Ils sont propriétaires d'une maison de famille ou disposent d'un pied-à-terre lorsqu'ils sont de passage en France ou quand leurs enfants viennent y faire leurs études.

Dès qu'ils quittent la France, leur résidence principale n'est plus qu'une résidence secondaire, qualification étonnante puisqu'il s'agit de leur unique résidence en France.

Aujourd'hui, nous examinons la proposition de loi de notre collègue Ronan Le Gleut, qui prévoit de faire de la résidence secondaire des Français de l'étranger une résidence d'attache et de les exonérer de la taxe d'habitation, sous certaines conditions. Sur le fond, je ne peux que partager les visées de la proposition de loi de notre collègue ; sur la forme, j'émets des réserves sur le dispositif retenu. Le texte ne crée pas, à mon sens, un statut distinct pour les biens détenus en France par les Français de l'étranger, il les classe dans une catégorie déjà existante, celle des résidences secondaires. Dès lors, introduire un traitement fiscal différent entre deux résidences secondaires, selon le lieu de vie de son propriétaire, soulève, selon moi, un risque d'inconstitutionnalité fort, qu'il faut à tout prix éviter. Le texte revu par la commission des finances ne prévoit le dégrèvement de la taxe d'habitation que pour les Français contraints de venir résider dans leur résidence d'attache en France pour des motifs extérieurs à leur volonté et pour assurer leur sécurité. Si cette exonération est la bienvenue, elle n'est que marginale. Elle n'est prévue que pour le temps que la situation se stabilise dans leur pays de résidence. Elle ne répond donc pas à la problématique de la résidence unique détenue par les Français de l'étranger. Avant d'envisager toute disposition fiscale particulière, il faut selon moi introduire une nouvelle notion en droit fiscal et créer une catégorie de résidence qui ne s'appuie ni sur la définition d'une résidence principale ni sur la notion de résidence secondaire.

Le bénéfice de la résidence « de repli », « d'attache » ou « intermittente »- le nom reste à trouver -pourra être conditionné soit à l'inscription des Français sur le registre consulaire, soit à la détention précédemment d'une résidence principale en France pour les personnes de nationalité étrangère qui y ont vécu et y conservent un bien.

Pour les Français de l'étranger, ce sujet n'est pas purement un problème fiscal : il est aussi symbolique et marque leur attachement inaliénable à la France. Dans tous les cas, je voterai pour cette proposition de loi, qui constitue une étape indispensable dans la construction d'un consensus parlementaire. Je reste convaincue qu'un nouveau statut conforme à la Constitution et au droit européen devrait être créé. La parole est

mais dont l'objectif est aussi partagé par ceux qui ne représentent pas les Français de l'étranger. Je ne rappellerai pas son objectif, le rapporteur et les auteurs de la proposition de loi l'ont déjà fait. à les remercier de leur idée judicieuse. Depuis de nombreuses années, nous évoquons le cas de nos compatriotes qui, par choix ou par obligation, se sont installés à l'étranger, pas forcément de

Que voulons-nous ? Que ces Français perdent totalement leur lien avec la France ? C'est ce à quoi s'emploie Bercy en estimant que leur domicile français est forcément une résidence secondaire,

fiscalité. Je regrette donc que le texte issu de la commission des finances contienne aussi peu d'avancées par rapport au texte initial. Selon moi, tout Français habitant à l'étranger devrait pouvoir qualifier sa résidence en France de « principale » et non de résidence « d'attache » ou « secondaire

le dégrèvement de la majoration sera limité à la seule année du retour sur le territoire et seulement en cas de danger dans le pays d'accueil. Je poserai deux questions.

que nous accueillions avec bienveillance l'esprit de cette proposition de loi puisque nous voulons créer, conformément à l'engagement du Président de la République, un statut de résidence de repli ou d'attache. J'ai néanmoins mis en avant les fragilités juridiques,

un dispositif fiscal. Dans la version initiale de l'article, il était prévu une exonération pleine et entière de la taxe d'habitation pendant toute la durée du séjour à l'étranger. L'amendement du rapporteur adopté en commission a

enceinte des forcenés de la fiscalité- plus on crée d'impôts, plus ils sont contents -et d'autres, dont je fais partie, qui souhaitent que la charge fiscale soit répartie de manière raisonnable et ne conduise pas

de la taxe d'habitation la résidence d'attache, qui est un logement vide, ne vise ni à interdire aux Françaises et aux Français qui vivent à l'étranger de garder leur résidence en France

déclaré comme résidence d'attache en France, sans avoir pour cela à payer une fiscalité supplémentaire. Nous nous sommes inscrits dans une logique par exception,

À titre personnel, pour l'avoir vécu directement, puisque j'y habite depuis vingt-six ans, je peux témoigner que, le 29 août 2005, un cyclone de catégorie 4 a frappé La Nouvelle-Orléans- ma maison s'est retrouvée sous 3 mètres d'eau,

revenant de pays classés en zone rouge par le ministère des affaires étrangères, là encore afin de tenir compte de situations très particulières plutôt que de créer un dispositif beaucoup trop général.

la représentation des élus des Français de l'étranger. De plus, il n'est donné à ce groupe de travail aucun ordre de mission précis. Cet amendement vise donc à dénommer ce groupe « commission » et, surtout, à en préciser la composition et les missions. Cette commission a vocation à être temporaire et le rapport contenant

Les Français établis hors de France font intégralement partie non seulement du destin national, mais également du dessein national. Le texte que nous allons- je l'espère ! -adopter aujourd'hui, par la création de cette résidence d'attache pour les Français établis hors de France, permet

Au-delà du pourtour méditerranéen et de l'Aquitaine, où nous assistons à une intensification de l'aléa incendie, nous constatons une extension de ce risque à de nouveaux territoires jusqu'alors épargnés. Cette évolution du risque a évidemment jeté une lumière particulière sur nos travaux et les a empreints d'une gravité et d'une urgence toutes particulières. L'examen de cette proposition de loi est l'occasion de démontrer les capacités d'anticipation et d'analyse du Sénat. Dans la suite de notre rapport d'information présenté en août 2022, nous nous étions fixé comme objectif initial de changer le droit avant la prochaine saison des feux. Il ne sera peut-être pas possible de respecter un tel délai, d'autant que- c'est un constat essentiel de notre rapport -la saison des feux commence de plus en plus tôt dans l'année. Pour preuve, depuis ce week-end, les Alpes-Maritimes sont déjà en train de brûler. Toutefois, l'aspect constructif de nos échanges avec les administrations centrales et déconcentrées et avec les établissements publics chargés de la forêt, l'engagement tout récent de la procédure accélérée

la proposition de loi est largement issue des contributions de ces mêmes acteurs à l'occasion de la conduite d'un premier cycle d'auditions au printemps 2022. Notre objectif étant d'aboutir au texte le plus robuste et le plus consensuel possible en vue de son inscription rapide à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale,

s'agit de tirer les leçons des retours d'expérience des feux, notamment après les épisodes dévastateurs qui ont embrasé la Provence en 2021 et la Gironde en juillet dernier.

notre stratégie de protection de la forêt et des espaces végétalisés repose sur deux piliers indissociablement liés : la préparation de la forêt à éviter le feu et, le cas échéant, à s'en défendre plus facilement,

bien qu'ils se distinguent par leur dimension économique respective. En effet, il apparaît que 1 euro investi au titre de la prévention et de la protection de la forêt préserve l'équivalent de 20 euros engagés lorsqu'elle est en feu. Cette approche en termes de « valeur du sauvé » souligne l'importance cruciale de la notion de défendabilité.

égard, nous avons réaffirmé la nécessité de faire figurer la protection des forêts contre l'incendie dans les documents de gestion durable des forêts, dans la stratégie nationale des aires protégées,

afin de procéder à des arbitrages relevant de l'intérêt général dès lors que l'on oppose- parce que l'on ne saurait pas les conjuguer - l'intérêt de la forêt à celui de la biodiversité. Il n'est pas acceptable que les acteurs de terrain soient entravés par des injonctions contradictoires, par exemple entre le code forestier et le code de l'environnement. L'objectif du législateur doit être de leur donner un cadre et des orientations clairs. Ensuite, nous devons poursuivre nos efforts pour assurer une application plus effective et plus complète des obligations légales de débroussaillement

C'est le signe du grand intérêt porté par le Sénat, chambre des territoires, à cette question cruciale, dont il s'était saisi avant même la saison des feux éprouvante de 2022. Je vous remercie de votre écoute et laisse sans plus tarder la parole à nos trois rapporteurs,

Nous avons parcouru un long chemin ensemble et nous espérons que le Gouvernement et l'Assemblée nationale permettront au texte de poursuivre sa route dans les meilleurs délais, car il y a urgence. J'aborderai, pour ma part, les articles dont j'avais la responsabilité au sein de la commission spéciale. Je commencerai par le titre I portant sur la stratégie nationale et territoriale pour renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie,

à la concertation en vue de définir la stratégie nationale et interministérielle. L'article 3 de la proposition de loi initiale ne faisait qu'encourager l'établissement d'un plan de protection des

Nous avons également complété le titre I par deux articles additionnels- les articles 7 et 7 -pour intégrer la stratégie nationale et interministérielle de lutte contre les incendies dans notre politique de gestion de l'eau et de protection de la biodiversité. Au sein du titre II visant à mieux réguler les interfaces forêt-zones urbaines, j'évoquerai les articles 12, 13 et 14 relatifs à l'intégration du risque incendie dans les politiques d'urbanisme. L'accueil ayant également été très positif

Au titre VI visant à sensibiliser les populations au risque incendie, deux principaux apports méritent l'attention : d'une part, afin de responsabiliser les fumeurs en milieu forestier,

particulièrement concernés par le travail engagé- je les salue et les remercie pour leur esprit de collaboration -, nous avons voulu tenir compte du retour d'expérience des feux qui ont durement frappé la Gironde l'année dernière, en donnant une assise juridique à la pratique des coupes tactiques.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, face à l'aggravation rapide du risque incendie et à la vulnérabilité grandissante des forêts, une part de la réponse réside dans une gestion active et concertée de la DFCI par massif. À cet effet, nous proposons de mobiliser les acteurs du monde forestier au sens large la gestion sylvicole comme levier de prévention et de défense des forêts contre les incendies. Une forêt non gérée est une forêt soumise à plus de risques : celui que le feu se développe avant d'être détecté, celui de ne pouvoir accéder au feu faute de dessertes aménagées et entretenues ou encore celui d'une progression rapide d'un incendie alimenté par une masse combustible. Pour répondre à ces risques croissants, nous proposons une stratégie à deux niveaux. Tout d'abord, nous entendons renforcer la prévention, en intégrant la prise en compte du risque incendie dans les documents-cadres de la politique forestière nationale. décliner et adapter localement cette stratégie aux réalités et aux pratiques de gestion durable et multifonctionnelle des massifs. Si elle représente des contraintes supplémentaires pour les propriétaires, les forestiers sont les premiers conscients de sa nécessité pour préserver leur forêt et sa biodiversité, ainsi que la production de matériaux.

nous préconisons des démarches collectives : mobilisation des acteurs locaux et singulièrement des élus, création d'associations syndicales de gestion ou de DFCI ... Par leur connaissance, leur veille attentive et leur gestion régulière des espaces naturels, ces acteurs sont déterminants dans l'efficacité de la stratégie de prévention et de lutte. Nous appréhendons la DFCI à l'échelle du massif forestier, plus pertinente pour que les acteurs s'approprient la politique de prévention en tenant compte des réalités territoriales de nos forêts, au-delà- et parfois en deçà -des limites administratives.

L'ensemble des dispositions proposées tirent les leçons des attaques sanitaires et des feux hors norme de 2022. Elles inscrivent dans le code forestier des principes généraux de diversification des essences et d'écoconditionnalité des reboisements appliqués par la plupart des gestionnaires forestiers, qui seront déclinés de manière opportune dans les documents-cadres régionaux. Voilà, mes chers collègues, les outils que nous proposons de mobiliser au profit des acteurs locaux pour une plus grande efficacité dans la prévention et la lutte contre les incendies. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme Jean Bacci, Anne-Catherine Loisier et Pascal Martin, c'est avec une grande satisfaction que je prends la parole devant vous pour vous présenter ce texte qui me tient particulièrement à coeur. J'aborderai les articles dont j'étais chargé au sein de la commission spéciale, en commençant par les obligations légales de débroussaillement, abordées au titre II. Si cet axe est tout à fait essentiel à la prévention des incendies, les OLD ne sont pourtant respectées qu'à hauteur de 30 %. elles évitent de mobiliser des moyens de lutte pour protéger les habitations et permettent donc aux pompiers de se concentrer sur la guerre contre le feu. Surtout, les OLD sont la meilleure garantie existante pour les particuliers les photos aériennes prises après l'incendie de Gonfaron, dans le Var, en 2021 montraient clairement que les propriétés de ceux qui avaient effectué un débroussaillement selon les normes n'avaient subi aucun dégât. Sur ce volet,

Par ailleurs, à l'article 11, nous avons souhaité rendre le dispositif plus robuste, en punissant pénalement ceux qui fournissent des attestations aux assurances faisant état de débroussaillements qui n'ont, en réalité, pas été réalisés.

en se mobilisant à l'été 2022, mettant à disposition leurs outils et leur force de travail dans la lutte contre les feux de forêt, en particulier en Gironde. Nous souhaitons, au travers de ce volet, les mettre à l'honneur : leur rôle, moins visible que celui d'autres acteurs, est tout aussi crucial dans la prévention.

À l'article 25, nous avons cherché à convaincre de la pertinence de notre dérogation à l'indemnité de défrichement dans les cas où celui-ci est réalisé dans un but de valorisation agricole ou pastorale renforçant la défense des forêts contre les incendies. cet article avait suscité des craintes et des plaintes : craintes des forestiers que des défrichements prennent prétexte de la DFCI et soient en fait abusifs ; plaintes du monde agricole, pour lequel l'indemnité de défrichement, même réduite de moitié, restait trop élevée pour être intéressante. nous avons encadré le dispositif par un décret et limité son champ aux seuls cas où un contrat engage l'exploitant à des coupures agricoles pérennes, ce qui permet de concilier les intérêts des mondes agricole et forestier. Il me semble que nous sommes parvenus à rassurer, rassurer, preuve que forestiers et agriculteurs peuvent travailler main dans la main pour prévenir ce risque, qui est de plus en plus intégré. La

les forêts nous rendent des services précieux, qu'ils soient économiques, en fournissant du bois-matériaux et du bois-énergie, ou environnementaux, en termes de biodiversité ou de stockage de carbone. En tant que ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, je rappelle que les forêts sont un véritable atout pour l'activité de nos territoires ruraux. Elles doivent donc être gérées et exploitées de manière durable pour continuer de fournir des services économiques et environnementaux à tous les Français. Mais elles doivent également être défendues face aux événements extérieurs. Les incendies hors norme de l'été 2022, provoqués par un concours de sécheresse et de températures particulièrement élevées, ont constitué une preuve éclatante et douloureuse des effets du changement climatique en matière de feux de forêt.

Les incendies ont toujours existé dans le sud de la France et reviennent malheureusement chaque été. Une politique volontariste de défense des forêts contre l'incendie a été mise en place dans les années 1980 et a produit de très bons résultats : les surfaces incendiées ont depuis été divisées par deux, voire par trois.

contre les incendies de forêt. Je veux notamment remercier chaleureusement, au nom du Gouvernement, les sapeurs-pompiers, les personnels de la sécurité civile, les sapeurs-sauveteurs, les forestiers sapeurs- en somme, tous les acteurs qui s'engagent pour la sauvegarde de nos forêts -pour l'excellent travail qu'ils effectuent au quotidien. quotidien. Le climat change : les incendies de l'été 2022 laissent entrevoir une intensification du risque dans les régions historiquement concernées- le Sud-Est, le Sud-Ouest, la Corse ... -, mais aussi et surtout une extension du risque dans des régions jusqu'ici préservées. Je pense notamment aux régions de l'ouest, de l'est et du centre de la France, territoires dans lesquels nous n'avions pas vu d'incendies de cette ampleur auparavant. Notre politique de défense des forêts contre l'incendie et de lutte contre ces incendies doit donc être renforcée et actualisée au regard d'un risque amplifié et étendu sur davantage de nos territoires.

Le rapport d'information publié en août dernier est de grande qualité et trouve aujourd'hui un écho dans cette proposition de loi. Cela traduit aussi l'engagement de longue date du Sénat à l'égard des enjeux forestiers, qui sont liés, naturellement, à la vie des collectivités territoriales, mais aussi, aussi, plus globalement, aux questions d'aménagement et d'avenir de nos territoires. Votre proposition de loi montre la diversité des politiques à conduire pour assurer la défense des forêts contre l'incendie. Ma présence devant vous aujourd'hui pour représenter le Gouvernement traduit le caractère multidimensionnel de ce sujet qui mobilise les compétences de trois ministères : le ministère de l'intérieur et des outre-mer, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Tout d'abord, la prévention est et demeure essentielle. Notre stratégie est d'éviter les départs de feux et d'être en mesure d'attaquer les feux naissants pour éviter leur propagation. Des moyens supplémentaires ont ainsi été accordés dès 2023 à l'Office national des forêts pour lui permettre de renforcer ses missions de surveillance et de première intervention et de les étendre dans les territoires nouvellement concernés par ce risque. des moyens supplémentaires ont été apportés par mon collègue Marc Fesneau à l'Association régionale de défense des forêts contre l'incendie (ARDFCI) des Landes de Gascogne, massif riche d'une organisation impliquant les propriétaires forestiers. Ce renfort de moyens se poursuivra en 2024.

et habitations. Soyons clairs, les obligations légales de débroussaillement fixées dans le code forestier doivent être mieux mises en oeuvre. En effet, lorsque leur mise en oeuvre est effective, les résultats parlent d'eux-mêmes. Avec Christophe Béchu et Gérald Darmanin, nous avons engagé des actions aux niveaux national et local pour sensibiliser le public concerné et accompagner les élus locaux, mais aussi pour sanctionner les négligences volontaires des propositions de simplification et de remobilisation des acteurs sont en cours de rédaction en vue d'une publication à l'été 2023, par voie réglementaire et à cadre législatif constant. constant. La proposition de loi examinée aujourd'hui permettra d'aller encore plus loin, en apportant des éléments de clarification, de simplification et de responsabilisation. Nos moyens de lutte doivent en effet être renforcés pour limiter la propagation des feux, protéger nos concitoyens et sécuriser nos infrastructures. Nous allons largement évoquer la prévention, qui est essentielle, mais pas suffisante. Malgré tout ce que l'on peut faire, le feu arrivera ; c'est pour cela que la lutte contre les incendies

d'y faire face dans les années à venir. Les conclusions de cette mission seront connues d'ici à cet été ; cela nous permettra de nous préparer pour l'année prochaine et les années suivantes. Cette proposition de loi loi est un signal fort envoyé aux propriétaires forestiers, aux riverains des forêts, aux associations de protection de l'environnement, aux élus locaux et à tous ceux qui agissent avec engagement au quotidien dans la prévention et la lutte contre les incendies de forêt. Il s'agit de leur montrer que nous sommes capables, ensemble, d'avancer pour nous adapter au changement climatique.

et interministérielle de défense des forêts contre l'incendie, qui permettra de mobiliser pleinement l'ensemble des acteurs, publics et privés, concernés. Vous proposez ensuite de faire évoluer la liste des territoires réputés comme particulièrement exposés aux risques d'incendie, ce qui constitue un moyen d'être réactif face aux évolutions du changement climatique. Le texte prévoit aussi d'améliorer l'articulation des mesures de DFCI avec d'autres politiques publiques, comme l'urbanisme et la protection des sites classés. Ainsi, nous serons collectivement plus à même de répondre au devoir de lisibilité pour les administrés.

également de la reprise dans la proposition de loi de deux évolutions issues de réflexions tenues par le passé dans le cadre des Assises de la forêt et du bois, à savoir l'abaissement à vingt hectares de l'obligation de disposer d'un plan simple de gestion et la systématisation de la télédéclaration.

L'attente de nos concitoyens porte en effet sur les incendies : c'est pourquoi nous souhaitons en rester principalement aux deux propositions, que nous trouvons équilibrées et qui sont issues du travail des rapporteurs et du passage du texte en commission. je souhaite saluer de nouveau la qualité du travail des auteurs de la proposition de loi et de la commission spéciale, et vous dire ma confiance sur le fait que nous pouvons enrichir ensemble ce texte afin d'assurer la cohérence et l'efficacité des mesures proposées, dont nous partageons les objectifs. La parole

Au total, 30 000 hectares de forêts sont partis en fumée en Gironde et plus de 60 000 hectares en France. Durant l'été 2022, la Gironde a brûlé d'un feu monstrueux, combattu avec abnégation par les pompiers dont je veux ici saluer le courage. Ces catastrophes, qui étaient jusqu'à présent exceptionnelles, seront demain la norme. En 2021 et 2022, nous avons connu les trois plus grands incendies de ces quarante dernières années

Des feux plus nombreux, plus étendus, plus violents : voilà à quoi nous devons nous préparer. De l'Aveyron à la Bretagne, en passant par la Gironde et les Vosges, après le Sud-Est, l'ensemble du territoire français est dorénavant concerné. Les experts sont unanimes : près de 50 % des forêts françaises seront menacées par le risque incendie d'ici à 2050. Malgré la mobilisation de deux mille sapeurs-pompiers, malgré les cinquante mille évacuations préventives et malgré la solidarité des milliers de bénévoles, les feux en Gironde ont souligné notre vulnérabilité au risque incendie. Nous devons en tirer les leçons. Je tiens à saluer le travail de la mission de contrôle et des rapporteurs qui sont à l'origine de cette proposition de loi. recommandations, le rapport d'information issu de cette mission a permis d'établir un diagnostic clair et partagé. Le texte que nous examinons aujourd'hui traduit l'essentiel de ces recommandations. Il permet, notamment, de renforcer les moyens des Sdis, de favoriser l'adaptation des forêts au changement climatique, de créer un nouveau droit de préemption pour les communes et d'établir des cartes d'aléas pour suivre l'évolution du risque. Après les feux gigantesques qui ont marqué l'été 2022, le Président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé une stratégie nouvelle de lutte et de prévention contre les incendies. Ce texte porte des mesures fortes. Il offre un début de réponse et ouvre la voie, mais il manque d'ambition sur plusieurs points essentiels. La prévention du risque incendie est la pierre angulaire d'une stratégie de long terme. Alors que 95 % des départs de feux sont d'origine humaine, acquérir une nouvelle culture du risque est un enjeu majeur. Les mesures proposées dans ce texte nous semblent insuffisantes. Nous déplorons également l'absence d'éléments sur le renforcement des moyens humains de l'ONF. Ses agents

De même, en pleine crise du volontariat et face à l'intensification du risque, il s'agira d'augmenter le nombre de sapeurs-pompiers professionnels et les moyens qui leur sont alloués. Notre politique de lutte contre les incendies doit tenir compte de l'évolution du risque sur l'ensemble du territoire. Cette stratégie passe par l'affectation équitable des moyens nationaux. Alors qu'un incendie doit être repéré et traité dès qu'il apparaît, la protection aérienne des Canadair et des Dash se révèle cruciale. Le temps d'autorisation et l'éloignement des appareils ne sont pas compatibles avec la temporalité des incendies. Il faut une flotte plus importante et une répartition adaptée de la flotte sur le territoire. Au regard de l'exposition colossale du sud-ouest de la France au risque incendie, un prépositionnement des moyens aériens, par exemple en Nouvelle-Aquitaine, paraît essentiel.

Enfin, nous restons vigilants sur les éventuelles dérives que le texte pourrait engendrer. La prévention et la lutte contre les incendies nécessitent des aménagements indispensables et des efforts importants. Mais elles ne peuvent se faire au détriment de la biodiversité et des écosystèmes, qui sont essentiels pour adapter nos forêts et réduire le risque. Permettez-moi, mes chers collègues, de citer Charles Darwin pour rappeler, ici, que « les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements ». L'équilibre à trouver n'est pas simple. Pour participer à ce rééquilibrage, sans jamais perdre de vue l'objectif de la proposition de loi, nous proposerons plusieurs amendements au cours des débats. Nous espérons qu'ils seront adoptés afin d'apporter des réponses à la hauteur des enjeux. Ce texte constitue néanmoins une première étape essentielle pour prévenir et lutter contre le risque incendie. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera pour cette proposition de loi. La parole

nous avons tous à l'esprit les images de l'été dernier, pendant lequel 72 000 hectares de nos forêts sont partis en fumée et avec eux autant d'hectares de notre patrimoine naturel. J'ai une pensée particulière pour mon département de la Drôme, où trente feux de forêt, dont celui de Romeyer dans mon Diois natal, ont brûlé 380 hectares et mobilisé plus de huit cents sapeurs-pompiers pendant dix jours.

avons heureusement pu compter sur le courage, l'efficacité et l'exceptionnel sens de l'engagement de nos forces de sécurité civile et des élus locaux. Je tiens ici à les saluer. Nous avons également pu compter sur l'aide de nos partenaires européens, avec l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne, permettant de mobiliser quatre avions de la flotte rescEU. Le caractère hors-norme de l'été 2022 ne doit pas cacher le fait que l'intensification des feux de forêt est un mouvement de fond : sur le pourtour méditerranéen français, les surfaces brûlées pourraient augmenter de 80 % d'ici à 2050. Les conséquences du changement climatique se manifestent de manière spectaculaire. Pour celles et ceux qui ne viennent pas de régions traditionnellement sujettes aux feux de forêt, l'été dernier a marqué un changement de paradigme, avec près d'un département sur deux concerné. À l'horizon 2050, 50 % des landes et des forêts métropolitaines seront exposées à un risque incendie élevé, contre un tiers il y a un peu plus d'une décennie. Cette extension est également temporelle, puisque la période à risque devrait être trois fois plus longue et que les feux hivernaux vont se multiplier. Dès le mois de mai 2022, le Sénat s'est saisi de ce sujet, puisque la commission des affaires économiques et celle de l'aménagement du territoire et du développement durable ont constitué une mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, mission à l'origine du texte que nous examinons aujourd'hui. Je veux ici remercier les rapporteurs qui l'ont élaboré. Les travaux de cette mission et de la commission spéciale ont mis en lumière le constat de la future vulnérabilité de notre stratégie de lutte contre les feux de forêt qui, bien qu'étant aujourd'hui un modèle en Europe, doit évoluer. Sans changement, notre stratégie ne suffira pas face à l'intensification et à l'extension des feux de forêt. La proposition de loi particulièrement dense qui a résulté des travaux de la mission répond pour partie à cette nouvelle problématique, en mettant l'accent sur l'aménagement du territoire, la gestion durable, la valorisation de la forêt et la mobilisation de l'ensemble des acteurs, au premier rang desquels les agriculteurs, maillons essentiels dans l'élaboration du modèle de lutte contre les feux de forêt au XXI siècle. Si, depuis 2017, nous avons investi de manière importante dans la sécurité civile, avec une augmentation budgétaire de 40 % et l'acquisition de nouveaux avions Dash, force est de constater que la mobilisation de moyens financiers est une condition nécessaire, mais insuffisante pour répondre à l'intensification de la pression qui s'exerce sur nos massifs forestiers. Au-delà des budgets, nous avons clarifié le cadre d'intervention des Sdis, conforté les plans communaux de sauvegarde et valorisé l'engagement et le volontariat lors de l'examen de la loi de Je retiens particulièrement la reconnaissance par la Nation du sacrifice ultime des sapeurs-pompiers, avec la création de la mention « Mort pour le service de la République » et la reconnaissance des enfants de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires décédés en service comme pupilles de la République. Nous sommes tous conscients que, si la France a un modèle de lutte contre les incendies performant et reconnu à travers le monde, nous devons néanmoins adapter nos politiques et nos territoires aux conséquences du dérèglement climatique. Autrement dit, il faut améliorer la prévention, renforcer les moyens de lutte et accélérer le reboisement post-incendie. Ce texte s'attelle à ces trois tâches et comporte un volet d'optimisation de la gestion de nos forêts que nos auditions ont mis en lumière comme étant un élément central du modèle à construire pour les années à venir. Le décloisonnement administratif qu'implique la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces boisées contre les incendies poursuit la logique d'optimisation de l'utilisation des ressources et d'assouplissement des procédures visant à renforcer la performance opérationnelle.

Nous instaurons un droit de préemption des parcelles de forêt sans document de gestion durable et présentant un enjeu au regard de la défense des forêts contre l'incendie, au profit des communes s'engageant à intégrer la parcelle au régime forestier. Nous renforçons l'application des obligations légales de débroussaillement. Nous conditionnons les aides d'État à des choix d'essences et de gestion adaptés au risque incendie. Nous reconnaissons, enfin, le rôle primordial des agriculteurs et de la sylviculture dans la prévention des feux de forêt. le texte permet donc de faire de la prévention, de lutter à la racine contre l'intensification et l'extension du risque d'incendie dans nos forêts, mais également d'adapter nos forêts et de conforter l'aménagement du territoire comme pierre angulaire de la protection de notre patrimoine naturel. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe RDPI votera ce texte. La parole

chers collègues, 72 000hectares ont brûlé en France en 2022, dont plus de 30 000 en Gironde, contre une moyenne de 8 500 hectares ces dix dernières années. Si le risque incendie avait, jusque-là, été globalement contenu par une politique volontariste de défense des forêts, les conséquences du réchauffement climatique changent totalement la donne.

arrive donc dans un contexte qu'on pourrait qualifier d'urgence. Nous saluons le travail transpartisan et collaboratif mené par les quatre mousquetaires, le président de la

avec une quinzaine d'amendements adoptés dès l'examen en commission, portant notamment sur : la prise en compte des spécificités organisationnelles des massifs forestiers et le rôle d'acteurs comme la DFCI là où elle est présente ; la prise en compte du risque incendie dans les documents d'urbanisme, même si ce qui est prévu ne nous semble pas encore suffisant ; l'instauration d'un congé spécial supplémentaire pour les sapeurs-pompiers volontaires ; la mise en place d'une communication spécifique aux propriétaires de terrains concernés par les OLD et l'augmentation du montant des amendes. Soulignons aussi que beaucoup de nos amendements ont été satisfaits par ceux des rapporteurs adoptés en commission, notamment : la reconnaissance législative des coupes tactiques et le caractère obligatoire

la réduction des cotisations patronales pour les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, une disposition que nous avions déjà proposée lors de l'examen de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile, dont le rapporteur était Patrick Kanner. De fait,

ascendante et non descendante ; la question de l'eau et du lien entre DFCI et plans de gestion en eau ; et l'amélioration de la connaissance des voies d'accès et des pistes DFCI avec un système de mise à jour de la cartographie.

L'État devra prendre ses responsabilités. Rappelons que les moyens humains et financiers tendent à baisser, aussi bien dans le domaine forestier que dans celui plus global de la prévention des risques- je rappelle que c'est au Sénat qu'on doit le « sauvetage » des moyens de l'ONF lors de la dernière discussion budgétaire.

Le Président de la République a présenté une « nouvelle stratégie » en octobre 2022- vous l'avez évoquée, madame la ministre -, mais nous attendons toujours une grande loi de programmation pour la forêt et une territorialisation des moyens aériens afin de lutter contre les feux hors norme, qui pourraient malheureusement devenir la norme. La

les incendies que nous avons connus l'été dernier ont détruit plus de soixante-six mille hectares de ce bien commun que sont nos forêts. La Gironde, les Bouches-du-Rhône, mais aussi la Bretagne : les incendies ont surpris par leur intensité, mais aussi par leur étendue géographique. Des forêts habituellement épargnées par les feux estivaux sont parties en fumée. Dans mon seul département, la Dordogne, ce sont deux cent quatre-vingts hectares qui ont été détruits. Ce qui semblait hier exceptionnel est donc en passe de devenir la norme. C'est ce que nous a rappelé la mission d'information sénatoriale constituée l'été dernier. En effet, les conclusions de cette mission pointent une intensification des feux en région méditerranéenne. Les surfaces brûlées pourraient augmenter de 80 % d'ici à 2050. Ces conclusions soulignent l'extension géographique du risque à des départements peu touchés et le développement d'incendies de végétation ou de terres agricoles. Pire, il n'y a plus de « saison des feux » ; la période à risque fort sera trois fois plus longue. Les incendies colossaux de l'été dernier nous rappellent que le changement climatique est déjà là, comme en atteste une fois encore le rapport du Giec. Ils ont mis en lumière la nécessité de penser de nouvelles stratégies d'adaptation pour la forêt et de renforcer les moyens de prévention et de lutte contre les incendies. Ils nous rappellent aussi que nos forêts sont fragiles. Outre le feu, la succession des sécheresses affaiblit les arbres, les rendant plus vulnérables aux attaques d'insectes et autres parasites. Nous assistons ainsi au dépérissement de certaines espèces. En ce sens, nous ne pouvons que saluer le travail effectué par les auteurs de cette proposition de loi qui nous rappellent la fragilité de ce patrimoine commun et la nécessité de le préserver. En effet, la stratégie française, qui a consisté à renforcer la prévention et la lutte contre les incendies et qui a permis durant des années de maîtriser la survenance de feux dits anormaux, est aujourd'hui bousculée par les changements climatiques. C'est pourquoi nous partageons la volonté de nos collègues rapporteurs d'anticiper le risque émergent, en l'intégrant de manière plus étendue dans les documents d'urbanisme et de planification des territoires jusque-là épargnés par les incendies de grande ampleur, ainsi que la prise en compte dans ces documents des espaces urbains, des terres agricoles et des massifs forestiers dans une logique de protection mutuelle. Nous saluons aussi le renforcement des OLD. La question des zones d'interface habitats-forêts est essentielle, car, dans ces espaces, le risque de départs de feux est élevé et la protection par les pompiers difficile et coûteuse. À cet égard, il serait opportun que les communes bénéficient de dispositifs d'accompagnement, y compris financiers. Nous partageons également la nécessité d'un renforcement de la sensibilisation des citoyens, élus et professionnels concernés. si les objectifs de ce texte sont louables et que les outils proposés sont pertinents, les moyens restent, encore une fois, insuffisants. Tous les acteurs que nous avons auditionnés l'ont dit : à moyens constants, il est impossible que les services de prévention puissent maintenir leur efficacité face à des feux de plus en plus intenses et fréquents. Comme le rappelait déjà le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, « le dérèglement climatique s'accélère. Il faut accroître le nombre de bombardiers d'eau, avions comme hélicoptères. Il faut aussi augmenter les moyens humains, et ce sans attendre ».

par la diversification des essences. Les forestiers doivent renouveler les peuplements dépérissants et adapter les forêts françaises en tenant compte des risques futurs. Il nous faut également renforcer les moyens humains et financiers face à l'intensification du risque incendie. Alors que la force de frappe des services d'incendie tient au maillage territorial, plus de deux mille sept cents centres d'incendie et de secours ont fermé ces vingt dernières années. Enfin, les difficultés à contenir les feux dans la région Sud-Ouest cet été nous ont rappelé le besoin d'une base aérienne de sécurité civile à l'ouest afin d'accroître la rapidité et l'intensité des interventions par Canadair. Par ailleurs, en trente-cinq ans, l'ONF, qui gère près de 25 % de la forêt métropolitaine, a perdu près de 40 % de ses effectifs. De seize mille salariés que comptait l'Office en 1986, il n'en reste plus que huit auxquels l'État continue pourtant de confier un nombre équivalent de missions et dont il exige une plus grande rentabilité. Les Sdis, l'ONF, le CNPF sont des acteurs publics garants de la résilience et de la résistance de la forêt. Ils doivent disposer des moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, qui- il faut le dire -se complexifient. Malgré ces réserves, nous voterons en faveur de cette proposition de loi.

Je viens de m'exprimer au futur, mais malheureusement il faut déjà parler au présent ... Les feux de forêt et de végétation sont plus graves d'année en année. Ceux de 2022 ont été dévastateurs, particulièrement en Gironde, mais mon département, le Morbihan, n'a pas été épargné non plus. Un incendie y a ravagé la légendaire forêt de Brocéliande. L'actualité espagnole nous rappelle cruellement cette urgence à agir : en six jours, le feu y a détruit la semaine dernière quatre mille trois cents hectares. Et nous ne sommes évidemment pas à l'abri de ce qui se passe sur la péninsule ibérique. Les feux sont de plus en plus nombreux et de plus en plus rapides, et la période de l'année durant laquelle le risque incendie est maximal s'allonge. Les chiffres avancés par nos rapporteurs, Anne-Catherine Loisier, Pascal Martin et Olivier Rietmann, dont je salue au passage l'implication et la qualité des travaux, sont éloquents : dans le Sud, les surfaces brûlées pourraient augmenter de 80 % d'ici à 2050. Les bois seraient progressivement remplacés par des maquis. D'ici au milieu du siècle, la moitié des landes et forêts métropolitaines seraient concernées par un risque incendie élevé, contre un tiers en 2010. Et la période à risque fort devrait être trois fois plus longue. D'où le mot du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France : « Aujourd'hui, la saison des feux, c'est toute l'année. » Il nous faut réagir, car nos dispositifs de lutte contre l'incendie commencent à ne plus être adaptés. Réagir, c'est ce qu'a fait le Sénat en constituant en mai dernier une mission de contrôle sur l'initiative de notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et de notre commission des affaires économiques. Je salue cette initiative au nom du groupe Union Centriste. La mission de contrôle a formulé un grand nombre de propositions. Nous nous réjouissons que celles d'entre elles qui relevaient de la loi aient été si rapidement concrétisées au sein du présent texte- c'est exemplaire De plus, l'approche opérée par le texte est extrêmement concrète, car elle est transversale. Elle articule prévention des feux et lutte contre l'incendie, ce qui constitue à nos yeux le seul moyen d'apporter une réponse véritablement efficace au problème posé. En allant de la stratégie nationale et territoriale au reboisement des parcelles brûlées, en passant par la promotion de la sylviculture, la sensibilisation des populations et l'équipement, le champ de la proposition de loi couvre l'ensemble des aspects générateurs du risque incendie. Le texte qui nous est aujourd'hui soumis est d'autant plus complet qu'il a été substantiellement enrichi par la commission spéciale, laquelle a tenu à tirer les leçons des feux de 2022 mettre en concordance la stratégie incendie avec les politiques de gestion de l'eau et de protection de la biodiversité et renforcer le caractère dissuasif des sanctions en cas d'absence de mise en oeuvre ou de non-respect des mesures de prévention et de lutte contre le risque incendie. L'un des aspects de cet enrichissement du texte nous tient particulièrement à coeur : il s'agit de la consécration du rôle préventif des forestiers et des agriculteurs. Nous ne remporterons cette guerre qu'avec leur appui. L'implication des communes est aussi essentielle, le rôle des élus locaux étant fondamental dans la politique forestière territoriale. En effet, si le maire est responsable de la sécurité sur son territoire, il a aussi un rôle essentiel de médiation dans la société et, de fait, la question forestière est devenue un sujet de préoccupation de nos concitoyens, au-delà des feux, dans de nombreux domaines : protection de la biodiversité, transition environnementale et énergétique. Ainsi, l'institution, à l'article 22, d'un droit de préemption pour les communes va dans le bon sens. Si une ou plusieurs parcelles sont identifiées comme étant stratégiques au regard de la défense de la forêt contre les incendies,

Je pourrais citer encore bien d'autres mesures essentielles comprises dans ce texte, mais vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera en sa faveur avec enthousiasme.

Sans attendre de nouveaux incendies dramatiques, mais sans oublier non plus les précédents, le Sénat, à la lumière des fameux « retex », les retours d'expérience, s'est donné les moyens de proposer une réponse d'envergure. Pour preuve, le texte tel qu'il ressort des travaux de la commission spéciale compte désormais plus de quarante articles et balaie ainsi l'ensemble des problématiques liées à la prévention du risque incendie dans nos territoires, à l'organisation de la défense contre le sinistre et à la gestion des massifs forestiers post-incendie. Pour reprendre une formule chère au président de notre groupe, Jean-Claude Requier, nous sommes face à un texte hétérogène, mais non hétéroclite. Cette hétérogénéité est un atout : la lutte contre l'embrasement se joue à de nombreux échelons. En oublier un risquerait de mettre en échec tous les autres. échelon est national. Dans votre rapport d'information du mois d'août dernier, madame, messieurs les rapporteurs, vous avez souligné très justement que « les politiques publiques de prévention et de lutte contre les incendies de forêt et de végétation se caractérisent par un portage politique et et administratif complexe ». Il est donc nécessaire d'oeuvrer à la mise en place d'une stratégie nationale et interministérielle, comme le vise le texte, aux fins de développer une approche transversale qui articulera à tous les niveaux de l'État la prévention contre les incendies et la sécurité civile.

Je me réjouis en ce sens de l'adoption par la commission spéciale de mon amendement qui vise à consulter les acteurs en charge de la défense de la forêt contre les incendies pour l'élaboration de documents d'urbanisme par les communes dont les bois et forêts sont classés et particulièrement exposés aux risques

Le texte y contribue, en tendant à financer des actions de communication afin de prévenir l'abandon de mégots ou bien en consacrant l'interdiction de fumer dans les forêts et bois classés à risque d'incendie. J'y vois de bonnes dispositions.

Cela étant, il reste encore de nombreuses améliorations possibles sur plusieurs points. J'y reviendrai lors de l'examen de mes amendements, pour beaucoup inspirés de ce que j'ai vécu et observé l'été dernier en Gironde.

cette proposition de loi signe une véritable prise de conscience. En effet, nous l'avons tristement constaté l'été dernier, désormais, c'est l'ensemble du territoire national qui peut être frappé par des incendies.

Au travers du texte qui est examiné aujourd'hui, il s'agit de traduire dans la loi certaines propositions de ce rapport sénatorial d'information, ce dont je me réjouis. En effet, pour m'être rendu sur le terrain et pour avoir échangé avec élus et membres du Sdis gardois, je sais à quel point

Conditionner la mutation d'un terrain concerné par les OLD au respect de ces dernières est une bonne chose, de même qu'accroître les sanctions administratives, mais aussi pénales, en cas de non-respect. Dans le même esprit, l'article 11, qui vise à rendre la franchise obligatoire dans les contrats d'assurance en cas de non-respect des OLD, a été enrichi pour punir pénalement les attestations aux assurances faisant état de faits matériellement inexacts. J'aurai pour ma part l'occasion de défendre un amendement qui vise à mieux informer les acquéreurs de parcelles concernées, notamment lors de leur passage devant le notaire, trop de maires regrettant encore que leurs administrés ignorent l'existence même de cette obligation. Il sera également question de l'indemnisation de ceux qui se substituent à leur voisin défaillant. L'article 13 de la présente proposition de loi dispose que l'autorité administrative compétente de l'État adresse aux communes une carte d'aléas permettant de cartographier, à l'échelle des communes concernées, les zones à risque d'incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation.

sont des prises de vues par satellite, avec leur lot d'erreurs, qu'il convient d'affiner en concertation avec les maires. J'ai en tête l'exemple de Fressac où le cimetière figurait en aléa feux très élevé ou d'autres communes qui ont dû notifier certaines erreurs manifestes, d'où l'importance, madame la ministre, de nourrir ce dialogue entre services de l'État et élus territoriaux. Pour toutes ces raisons et d'autres encore qui seront évoquées par mes collègues, je voterai, comme mon groupe, cette proposition de loi. Elle va dans le bon sens,

! Permettez-moi de rappeler- nous sommes nombreux ici à le savoir -que ce sont presque toujours les communes rurales, petites par leur démographie, mais très grandes par leur surface, qui doivent faire face à ces feux. Les élus de ces communes n'attendent pas que Paris leur indique quoi faire, mais que des moyens supplémentaires leur soient alloués, par exemple pour rénover leurs bornes incendie, embaucher de jeunes surveillants durant l'été, installer des bâches à eau ou financer leur propre débroussaillement. Pour conclure, nous ne pouvons plus nous contenter de déplorer les effets dont nous chérissons les causes. Nous devons nous adapter au réchauffement climatique, mais aussi accélérer notre transition écologique, notamment, madame la ministre, en facilitant l'accès au fonds vert pour nos communes rurales. Mes chers collègues, nous sommes désormais en 2023, nos forêts brûlent et nous ne pouvons plus regarder ailleurs ! La parole

Ce dispositif est l'alliance de beaucoup de choses en lesquelles je crois et qui font la différence : l'association des efforts publics et privés, la vision d'une écologie libérale, une gestion durable qui allie

Je salue tous les membres de la commission spéciale qui ont eu à coeur de faire de ce texte la réponse aux nombreuses problématiques que nous rencontrons. Je tiens tout particulièrement à souligner le travail de nos rapporteurs, à l'écoute et investis. Nos objectifs sont clairs : tirer les leçons des derniers mois

Une gestion durable et équilibrée est la clé de la résilience. Parce que la forêt est un lieu extraordinaire, les problématiques auxquelles elle fait face le sont tout autant. Les solutions apportées dans ce texte ouvrent la voie aux évolutions que nous devons déployer. De manière générale, il faut inclure systématiquement le risque d'incendie dans les documents d'urbanisme. À cet égard, la gestion durable de la forêt paraît relever du bon sens ; permettre une évolution et donc prévoir de la souplesse dans les documents et stratégies le sont tout autant. La prévention est la base de l'adaptation. Quand il s'agit de lutter contre le risque d'incendie, cette affirmation prend tout son plus, les bons financements et la mise à disposition de moyens seront cruciaux dans les mois et années qui arrivent. À ce titre, je vois la pérennisation du Defi forêt comme une bonne nouvelle. Son encadrement me semble pertinent : les bonnes pratiques sylvicoles sont encouragées, elles méritent d'être accompagnées.

et leur en donner les moyens est crucial. Chacun sait la complexité du morcellement et l'enjeu que cela représente en matière de capacité de gestion. Je salue particulièrement les agriculteurs et leurs actions déterminantes l'été

les communes, point de lutte contre les incendies. Dans l'Aude, soumis depuis des décennies aux incendies ravageurs, nous savons qu'elles sont essentielles. Elles créent et entretiennent les équipements indispensables aux pompiers dans la lutte contre les feux : pistes, citernes, zones d'appui, etc. Cela représente- vous le savez -des investissements qui pèsent lourdement sur les finances communales. communales. En Occitanie, les communes n'ont d'ailleurs pas attendu les ordres venus d'en haut pour investir dans la prévention et dans les moyens de lutte, et ce depuis plus d'un demi-siècle. Les communes sont indispensables. Avec leurs groupements, elles consacrent des budgets de plus en plus importants à la mise en oeuvre des politiques de défense de la forêt contre les incendies, au travers notamment du financement des services départementaux d'incendie et de secours. Les communes sont primordiales, car les maires, dans le cadre du pouvoir de police que leur a délégué l'État, sont en pleine responsabilité sur ces sujets, dont ils sont d'ailleurs pénalement responsables.

il faut associer pleinement les élus des communes, notamment forestières, à la définition des politiques de prévention et de lutte contre l'incendie.

Enfin, il faut adapter les dispositifs aux enjeux contemporains. Mes chers collègues, la proposition de loi qui nous réunit cet après-midi est le fruit d'un travail important qu'il convient de saluer. Il était urgent d'élargir la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les incendies, en intégrant la prévention et la lutte dans les documents d'urbanisme et dans les différentes missions des opérateurs de l'État. Il faut accompagner les particuliers et le monde agricole dans le respect et la mise en oeuvre de leurs OLD. Toutefois, je me permettrai de souligner plusieurs écueils. D'abord, comme ma collègue Laurence Harribey l'a souligné, l'État doit être à la hauteur des enjeux financiers. Ensuite, nous estimons qu'il est important de véritablement placer les élus des communes forestières au coeur des dispositifs, parce qu'ils sont incontournables et constituent le pivot des politiques de prévention et de lutte contre les incendies.

dans un souci de simplification et d'efficacité des dispositifs, nous avons souhaité, lorsque nous avons examiné le titre II de ce texte, la création d'un diagnostic des obligations légales de débroussaillement sur le modèle du diagnostic de performance énergétique. Un tel diagnostic, d'une part, renforcerait

Enfin, nous pensons que la mobilisation contre le risque incendie doit concerner l'ensemble des acteurs de la société, y compris les plus jeunes. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'ensemble de ces éléments au cours de l'examen de ce texte. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « des incendies dévoraient le ciel aux quatre coins de l'horizon », « les nuits n'étaient plus noires, mais rouges » : ces mots

d'autant plus que la sécheresse hivernale actuelle laisse présager de nouveaux records d'incendies. Baisserons-nous les bras pour autant ? Non L'intensification des feux de forêt n'est pas une fatalité et le travail méticuleux des auteurs et des rapporteurs de cette proposition de loi redonne volonté et espoir à ceux qui combattent le feu, à commencer par nos pompiers. Dans cette lutte, ils ne sont pas seuls, et je veux d'abord souligner le rôle fondamental des collectivités territoriales. Les plans de prévention des risques d'incendies de forêt (PPRIF) constituent un bon outil et je soutiens la volonté d'encourager les collectivités à se regrouper selon une logique de massif. En effet, le feu ne s'arrête pas aux frontières communales. Je salue la création, à laquelle tend cette proposition de loi, d'une délégation à la protection de la forêt inspirée d'une structure associant déjà les départements méditerranéens, ainsi que la Drôme et l'Ardèche, et dont je peux témoigner de l'utilité. Nous devons, à tous les niveaux, faciliter l'action de ceux qui combattent le feu en première ligne : les pompiers de nos Sdis. Comme le préconisent nos rapporteurs, il faut faire respecter beaucoup plus strictement les obligations légales de débroussaillement. C'est un point crucial, car le défaut de débroussaillage provoque des feux en zone habitée qui pourraient être évités. En cela, ils concentrent les efforts de nos pompiers et les détournent de la stratégie générale de lutte contre les sinistres.

Je pense notamment aux cultures faisant office de coupe-feu, comme les oliveraies ou les vignes entretenues. Suivant cette logique, le réaménagement effectué à la suite d'un incendie de forêt est primordial. Il s'agit non seulement de réhabiliter les espaces détruits, mais également de les aménager de telle sorte qu'un futur feu verra ses effets amoindris. Il faut enfin parer à l'apparition d'autres risques, comme les glissements de terrain survenant à cause de la perte du couvert végétal. Je veux rappeler ici que la force menante contre les incendies, ce sont les Sdis. À ce sujet, je me félicite de l'opiniâtreté de nos rapporteurs qui ont introduit des dispositions déjà promues par le Sénat, à savoir la réduction des cotisations patronales pour les employeurs de pompiers volontaires et la suppression de la TICPE pour les Sdis. Dans leur lutte contre des feux dévorants extrêmement violents, comment imaginer que nos services de secours puissent être empêchés ici par une pénurie de matériel, là par un problème de personnel ou de formation ? Sans un appui financier plus prononcé de l'État, leur engagement sera difficilement supportable. L'été 2022 nous en offre la plus dramatique illustration, avec des Sdis à la limite de la rupture. Une politique publique de lutte contre les incendies est extrêmement coûteuse et concerne autant l'État, les collectivités, les agriculteurs, les services de secours et les particuliers. Nous savons que les décennies à venir seront plus chaudes, que les feux seront plus fréquents et sur des périodes de l'année plus étendues. Anticipons, madame la ministre, et lançons une stratégie sur le long terme avec des plans de financement pluriannuels conclure, je tenais à saluer et à encourager les réserves citoyennes de sécurité civile, comme celle récemment créée à Lagorce, dans mon département, l'Ardèche. Elles ont pour mission d'agir en amont, de patrouiller et d'aider les pompiers. En accompagnant les soldats du feu et en complétant les efforts importants fournis par les agriculteurs, elles permettent aux citoyens de s'engager eux-mêmes clans la défense de leur environnement, montrant ainsi que les ravages ne sont pas inéluctables. La parole

tant en matière de surface brûlée que d'émissions de carbone : plus de 785 000 hectares sont partis en fumée du 1 janvier au 19 novembre. C'est plus du double de la moyenne de 317 000 hectares brûlés annuellement entre 2006 et 2021. Ces incendies ont entraîné des émissions totales de carbone pour 2022 estimées à 9 mégatonnes,

c'est l'un des trois départements soumis au plus fort risque d'incendie de forêt dans la région méditerranéenne. Permettez-moi, mes chers collègues, de saluer le sang-froid de l'ensemble des maires qui font face chaque année à des incendies bien souvent criminels. Je me souviens du feu de la Montagnette l'été dernier dans le nord du département et des incendies qui ont ravagé les Calanques à diverses reprises,

Anne-Catherine Loisier, Pascal Martin et Olivier Rietmann ont ainsi fait un travail remarquable en nous présentant aujourd'hui un texte qui comprend trente-huit mesures. Nous ne réussirons pas cette lutte contre les incendies sans sensibiliser la population. feux sur dix sont d'origine humaine et sept sur dix seraient liés à l'imprudence humaine. Aussi, toute utilisation du feu peut être source de départ d'un incendie de forêt. C'est pour cette raison qu'une attitude citoyenne et la vigilance de chacun sont impératives. L'information et la sensibilisation sont indispensables. L'article 30 prévoit de s'appuyer sur la filière de responsabilité élargie du producteur, la REP, pour financer des actions de communication afin de prévenir l'abandon de mégots, notamment dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie et dans les bois et forêts classés à risque d'incendie. Nous ne réussirons pas sans sanctions. C'est pourquoi l'article 31 a pour objet de consacrer au niveau législatif l'interdiction de fumer dans un bois ou une forêt classée à risque d'incendie. Enfin, mes chers collègues, je ne pouvais prendre la parole aujourd'hui sans rendre un hommage appuyé à l'ensemble des pompiers. Non sans un certain chauvinisme, que j'assume, je veux saluer l'engagement des marins-pompiers de Marseille et du Sdis des Bouches-du-Rhône. Est-il plus noble et plus belle mission que celle qui consiste à risquer sa vie pour en sauver d'autres ? S'il est une famille unanimement aimée et respectée, qui force l'admiration de tous, en France, c'est bien celle que forment les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers. Je crois qu'unanimement nous pouvons leur dire merci ! Ce texte consacre son titre VII- articles 32 à 34

mesure phare, il s'agit d'instaurer une réduction de cotisations patronales pour les entreprises et administrations, en contrepartie de la disponibilité de leurs employés et agents exerçant en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Aussi, je dis à nos pompiers qui suivent nos débats : les Français savent tout ce que votre mission représente d'engagement et de sacrifice ; ils savent que vous la remplissez avec tout votre coeur, toute votre intelligence et tout votre talent. Soyez-en remerciés, parce que c'est vous qui préservez nos vies, notre patrimoine et nos paysages ! La discussion

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, alors que notre pays a été confronté l'été dernier à des feux de forêt d'une intensité rarement égalée, je me félicite que notre assemblée se saisisse de cette problématique. À cet égard, je tiens à saluer le travail des auteurs de ce texte. Le texte que nous étudions aujourd'hui a pour ambition première d'adapter les outils de lutte et de prévention aux nouveaux défis du changement climatique et, plus particulièrement, à la vulnérabilité grandissante des massifs forestiers. Ce risque s'étend à des territoires jusqu'alors épargnés. Je voudrais évoquer le cas particulier de mon département de la Meuse et de sa zone rouge qui représente douze mille hectares du champ de bataille de Verdun, où le sol est d'une est d'une nature toute particulière. En effet, il renferme nombre de munitions et d'obus présentant encore une grande dangerosité. Sur ce sol, le risque incendie est particulièrement prégnant. Il a d'ailleurs été renforcé par les attaques de scolytes et le dépérissement- cette forêt est composée en partie de résineux. Nous sommes obligés de le constater, en cas de gros incendie, une intervention à pied n'est pas envisageable. Il est donc absolument indispensable de renforcer la prévention, la coordination et les moyens d'intervention, notamment aériens. Enfin, ce texte vise à améliorer l'aménagement et la valorisation des forêts, en appréhendant la DFCI à l'échelle de chaque massif forestier. Il permet donc une prise en compte spécifique des territoires. La parole est à M.

l'article 1 de la proposition de loi porte sur la stratégie nationale et territoriale permettant de renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Cet article prévoit plus particulièrement l'élaboration d'une stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts contre l'incendie. Il s'agit donc de faire collaborer encore mieux les ministères chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, en concertation avec l'ensemble des représentants des professionnels chargés des missions de sécurité civile. À ce titre, il convient de rappeler les engagements du Président de la République formulés lors de son allocution du 28 octobre 2022 à la suite des terribles incendies de Gironde. Parmi ces engagements, j'ai relevé la création d'une quatrième unité militaire d'instruction et d'intervention de la sécurité civile d'ici à 2024. Cette unité serait créée dans le sud-ouest de la France,

Elles sont la fierté de la France et portent secours aux sinistrés en cas d'événements climatiques, tremblements de terre et autres catastrophes. 2024, c'est demain : la création, dans la précipitation, de cette unité pourrait avoir un impact dommageable sur les moyens et sur les ressources humaines des trois unités existantes. J'ai récemment visité l'unité d'instruction et d'intervention de sécurité civile n° 7 de Brignoles, dont j'ai pu apprécier le niveau d'équipements, le professionnalisme, ainsi que les qualités humaines des femmes et des hommes qui y travaillent. La complémentarité de leurs missions avec celles des sapeurs-pompiers de nos départements nécessite de créer au plus tôt cette quatrième unité, améliorant ainsi la stratégie nationale. Nous ne pouvions

Il faut changer de regard sur le risque incendie. Les incendies, qui sont, à plus de 90 %, d'origine humaine, involontaire ou non, sont aujourd'hui d'une telle

Après l'été 2022, à la rentrée de septembre, j'avais pris l'initiative de proposer au ministre de l'intérieur de décerner une agrafe « Feux de forêt 2022 » aux sapeurs-pompiers qui avaient été mobilisés pendant tout l'été, ainsi qu'aux bénévoles des comités communaux des feux de forêt.

J'avais adressé un courrier en ce sens le 21 septembre au ministre de l'intérieur. Le jour même, lors d'une audition de la commission des lois, je l'avais interrogé sur cette initiative. Il m'avait dit qu'il y souscrivait et qu'il donnerait une réponse favorable dans les meilleurs délais.

Gisèle Jourda. Cet amendement vise à préciser la liste des personnes morales ou structures qui seront associées à l'élaboration de la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies. Il s'agit d'inscrire explicitement dans la loi la présence des communes forestières dans ce travail de concertation. Ces dernières sont en effet incontournables en matière de gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques. Elles constituent à ce titre le pivot d'une politique de prévention et de lutte contre l'incendie efficace sur nos territoires. La rédaction actuelle de l'article 1 pourrait donner le sentiment que notre amendement est satisfait, puisqu'il prévoit la présence des collectivités territoriales et de leurs groupements. Or nous pensons que la loi se doit d'être précise dans un certain nombre de cas afin de lever tous les doutes possibles. Ainsi, lorsqu'il est question de notre stratégie nationale de lutte contre les incendies, la place des communes forestières doit être considérée à part entière et reconnue comme telle dans la loi. Nous estimons également que la liste des personnes associées à l'élaboration de la stratégie nationale prévue à l'article 1 étant déjà importante, cet amendement ne rendra pas la loi plus bavarde, tout en ayant le mérite de la clarté.

Cette stratégie sera le fruit d'une collaboration entre de nombreux acteurs, parmi lesquels les ministères chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile des représentants des acteurs de la sécurité civile, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles, ainsi que des organisations de protection de l'environnement.

Cet amendement vise à inclure les chambres d'agriculture dans l'élaboration de la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies.

dans l'élaboration de la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies. En effet, les chambres d'agriculture, de par leur connaissance des enjeux de la prévention et de la lutte contre les incendies dans les espaces agricoles comme boisés, sont des acteurs

la concertation à d'autres structures agricoles. Si les chambres d'agriculture ont leur place dans la concertation sur cette stratégie, nous souhaitons aller plus loin, en associant d'autres organisations professionnelles agricoles, notamment les représentants du pastoralisme. Le pastoralisme peut en effet jouer un rôle essentiel pour la gestion du risque incendie. Le rapport d'information sénatorial dont est issue cette proposition de loi a bien montré les synergies possibles. Il existe différents outils développés par les acteurs locaux, comme le partenariat entre l'ONF et des agriculteurs pour mettre en oeuvre le pastoralisme sur les territoires à risque.

Elles permettent de maîtriser l'embroussaillement et la présence d'un sous-étage inflammable, d'entretenir des coupures de combustible ou de constituer des mosaïques entre milieux ouverts et milieux forestiers. Les acteurs des systèmes agricoles pastoraux sont demandeurs. Ils souhaitent être associés à la politique de lutte contre les risques d'incendie. Nous pensons que la concertation et le dialogue sont une partie de la solution. Mettre tous les acteurs autour de la table nous paraît essentiel. Quel est l'avis

de trouver les voies et moyens pour concilier protection de la biodiversité et prévention des incendies. Dès lors, il n'y a pas lieu de limiter la participation à cette concertation aux seules ONG environnementales dont l'objet est en lien avec la prévention et la lutte contre les incendies. Si cet amendement était adopté, il est même possible qu'aucune ONG ne soit en état de participer à cette concertation, car il est probable qu'aucune ne réponde à la définition proposée.

En accompagnement de la simplification proposée par l'article 2 visant à classer les massifs à risque d'incendie par arrêté ministériel pour avoir plus de souplesse et de réactivité par rapport à l'évolution de ce risque, il doit être mis en oeuvre une méthodologie homogène au niveau national permettant ce classement. De même, il est important de préciser les consultations locales qui doivent être réalisées au niveau départemental classement., celui-ci servira de base pour définir la réglementation départementale à appliquer en matière de DFCI- emploi du feu, pénétration dans les massifs et réglementation des activités. C'est la raison pour laquelle cette nouvelle procédure doit faire l'objet, selon nous, d'un cadrage par décret. Quel est l'avis de la commission

Au regard de l'augmentation du risque incendie et de son évolution géographique, nous nous accordons sur cette nécessité et nous jugeons cette proposition pertinente. Toutefois, nous souhaiterions que la voix de nos territoires puisse également être entendue. C'est pourquoi nous proposons de donner la possibilité aux territoires, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, de faire part, par la voix du président du conseil départemental, de leur souhait de figurer parmi les territoires particulièrement exposés au risque incendie. Cet amendement tend donc à instaurer une logique montante, et non pas exclusivement descendante, pour laisser aux élus, qui sont en première ligne et qui savent mieux que quiconque

sur le classement des bois et forêts « à risque ». L'amendement est donc satisfait sur ce point. En tout état de cause, la formulation de l'amendement pose problème : le classement « à risque » porte sur les bois et forêts

il a été déclaré irrecevable au motif qu'il était satisfait par l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent,

et groupements peuvent donc déjà émettre un avis défavorable sur un PPFCI : sur ce point, l'amendement proposé est satisfait. L'objet de l'amendement précise que l'intention de ses auteurs est de rendre cet avis conforme.

je ne suis pas certain de la pertinence d'un passage à un avis conforme. D'une part, une telle demande ne nous a jamais été formulée par les associations de collectivités, notamment par la Fédération nationale des communes forestières part, nous ne souhaitons pas alourdir les processus d'adoption des documents stratégiques de prévention incendie. Notre objectif est même d'alléger leur élaboration et leur mise à jour.

Les sénateurs du groupe SER estiment qu'au vu de la récurrence des incendies, de leur intensification et de leur extension sur l'ensemble de notre territoire ce délai de cinq ans est trop important pour permettre permettre une réactivité suffisante face à la forte évolution de ce risque. Nous proposons une solution plus adaptée, avec une évaluation au moins tous les trois ans. Ce nouveau délai permettrait,

que cette évaluation donnera nécessairement lieu à des modifications : elle ouvre seulement une possibilité.

Il ne me semble pas pertinent de passer à trois ans, comme tend à le prévoir cet amendement, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la durée d'un PPFCI est au plus de dix ans : notre idée est donc d'avoir une évaluation du plan à mi-parcours. ailleurs, nous souhaitons orienter les acteurs vers une démarche d'évaluation régulière, sans les contraindre à appliquer le même modèle partout sur l'ensemble du territoire. Notre rédaction précise que cette évaluation s'effectuera « au au moins » tous les cinq ans : si la réalité locale nécessite une évaluation plus récurrente, ce sera donc tout à fait possible. Laissons aux acteurs locaux le soin de définir les modalités de mise en oeuvre des PPFCI les plus pertinentes en fonction des réalités territoriales

paraît être un rythme très difficile à tenir pour les acteurs. Rien n'empêche, si les circonstances le méritent, qu'un plan soit évalué au bout de trois ans, mais contraindre tous les départements à s'astreindre à un tel exercice nous semble inutilement chronophage. Madame

Les événements survenus pendant l'été 2022 nous auront démontré la nécessité de renforcer notre politique de prévention contre les incendies, mais également d'améliorer l'articulation entre les différents acteurs qui sont amenés, en cas de crise, à intervenir sur le terrain.

permettant à ses acteurs de tirer les enseignements des événements passés et de partager leurs expériences et leurs ressentis une analyse. Ce retour d'expérience, ou retex comme certains l'appellent, se pratique déjà dans de nombreux domaines, sanitaires ou industriels. Par cet amendement, nous souhaitons le développer en matière de lutte contre les incendies.

qu'il en soit, cela relève non pas de la loi, mais des compétences générales et du pilotage du préfet. Comme vous le soulignez, c'est au préfet d'organiser en interministériel et avec les acteurs du territoire ce retour d'expérience. Par ailleurs, la liste des participants que vous

de Deci à un syndicat forestier ou à un groupement de collectivités compétent en matière de réglementation de défense extérieure contre l'incendie.

d'ouvrir la possibilité de transfert de la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie vers les syndicats des eaux qui sont déjà dotés de la compétence de défense extérieure contre l'incendie.

a fait l'objet d'un travail d'ensemble sur la compétence Deci de la part nos collègues de la commission des lois. Il convient d'en maintenir la cohérence dans un texte dédié. C'est pourquoi, sans me prononcer sur le fond de ces deux amendements, j'émettrai un avis défavorable afin d'éviter d'alourdir la navette parlementaire avec des dispositions redondantes.

spéciale. L'amendement n° 56 vise à étendre la possibilité de transfert de la police spéciale de la Deci au président des groupements compétents en matière de Deci après accord unanime des maires concernés. Nous ne sommes pas opposés à un tel transfert, dès lors que celui-ci est conditionné par le fait que le groupement dispose de la compétence en matière de Deci. Cependant, la condition d'unanimité remet en cause les dispositions applicables au transfert facultatif de police spéciale dans le cas des communautés urbaines. Afin de ne pas multiplier les mécanismes de transfert, le Gouvernement n'est pas favorable à la fixation d'une condition générale

plans, schémas, etc. -de lutte contre les incendies dans les documents d'urbanisme. C'est d'ailleurs l'objet plus général de cette proposition de loi qui, au travers de nombreux articles, s'inscrit totalement dans cette volonté.

L'amendement n° 62 s'inscrit dans une logique similaire. Il vise à ce que le schéma communal de défense extérieure contre les incendies et le plan local d'urbanisme ou la carte communale soient cohérents grâce à la prise en compte de la Deci dans l'élaboration des documents d'urbanisme. Nous proposons ainsi de compléter l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, qui liste actuellement les schémas,

l'élaboration d'un schéma communal de défense extérieure contre l'incendie est facultative. Sa prise en compte explicite par les plans locaux d'urbanisme, comme vous le proposez,

chargée de l'animation et de la coordination des services de l'État en matière de défense des forêts contre les incendies. Afin d'éviter que les missions de cette délégation empiètent sur d'autres services existants, il convient de limiter son champ d'intervention aux seules missions d'animation et de coordination. Quel est l'avis de la

n'emploie que quatre personnes : difficile dans ce cadre d'empiéter sur les compétences des autres services de l'État. Par conséquent, l'avis est défavorable sur cet amendement

des services de l'État. L'organisation des services de l'État, que ce soit au niveau national ou territorial, relève de la compétence réglementaire et non du législateur. À l'échelon déconcentré, comme c'est le cas ici, il revient déjà aux préfets d'assurer la coordination

présenter l'amendement n° 25 rectifié. L'article 6, dans sa rédaction actuelle, prévoit qu'en fonction des circonstances locales pourrait être établie, sous l'autorité de chaque préfet de zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt chargée de l'animation et de la coordination des services de l'État en matière de défense des forêts contre les incendies. Sur ce sujet, il est impératif de favoriser un travail interservices n'oubliant aucun acteur local.

Ainsi, dans une recherche d'efficacité et d'économies, la constitution d'une telle délégation en Nouvelle-Aquitaine devrait associer impérativement la Fédération régionale des associations syndicales autorisées, dès lors qu'il en existe une. Le Sénat est à même de comprendre la nécessité de s'adapter et d'intégrer les solutions locales, quand elles ont fait leurs preuves, de ne pas empêcher le préfet de s'adapter à son écosystème local. La parole l'amendement n° 33 rectifié. Depuis de nombreuses années, l'organisation locale dans le Sud-Ouest favorise le travail interservices de manière informelle au sein de la Fédération régionale des ASA de DFCI, avec des habitudes de travail bien établies.

Il paraît donc utile d'associer les fédérations régionales des ASA de DFCI, dans les territoires où elles existent, à ces nouvelles délégations de protection de la forêt.

que la création d'une délégation à la protection de la forêt ne signifie pas la fin des associations de DFCI : ces deux réseaux, qui n'ont pas les mêmes finalités, seraient au contraire complémentaires et participeraient en commun à la prévention des incendies de forêt. Les associations de DFCI, pour utiles et nécessaires qu'elles soient, sont des associations qui réunissent les propriétaires forestiers. Elles n'ont donc pas le rôle de coordination des divers services déconcentrés que nous souhaitons voir mis en place. En effet, l'objectif des délégations à la protection de la forêt est non pas de constituer une nouvelle entité qui serait composée de l'ensemble des acteurs de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt, publics comme privés, la rendrait rapidement inopérante, mais de favoriser l'interministérialité au sein des services déconcentrés de l'État à travers une structure dédiée, disposant de moyens humains et financiers propres. L'instance de dialogue entre tous les acteurs de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt trouve sa place non pas dans la délégation à la protection de la forêt, mais dans la définition de la stratégie nationale et interministérielle que nous venons de voter à l'article à l'article 1. C'est pourquoi je ne suis pas favorable à vos amendements, dont la première phrase aurait pour conséquence de détricoter la mesure que nous portons, tandis que la seconde est superfétatoire dans la mesure où la Fédération régionale des ASA de DFCI d'Aquitaine- c'est elle qui est concernée -est déjà partenaire de l'État et de la préfecture de région.

entraînerait en sus la création d'une nouvelle catégorie de structures administratives. Le Gouvernement souhaite que, sous l'égide des préfets, la gouvernance locale des acteurs soit effective en matière de prévention et d'action de lutte contre les feux de forêt sans qu'il soit besoin de passer par le vecteur législatif. Cela existe déjà dans les territoires qui connaissent des épisodes de feu depuis plusieurs années, et cela sera le cas dans tout territoire qui, à cause du changement climatique, sera demain soumis à un risque de feux de forêt. Je vous demande donc de bien vouloir retirer ces deux amendements, faute de quoi l'avis du Gouvernement sera défavorable. Madame

est à Mme Laurence Harribey. Cet article 7 vise à intégrer dans les objectifs de la recherche appliquée sur la forêt et le bois un objectif d'adaptation au changement climatique, à la promotion de pratiques et itinéraires sylvicoles, qu'à la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. En commission spéciale, une dimension supplémentaire a été introduite afin que les risques associés au changement climatique soient également pris en compte, ce dont nous nous félicitons. Cet amendement vise, quant à lui, à préciser explicitement que cette recherche d'adaptation et de résilience doit également passer par une recherche accrue sur les bénéfices induits par une diversification des essences dans les politiques de replantation. Nous avons bien conscience que les chercheurs ont déjà à l'esprit cette dimension, mais cet article ayant vocation à préciser le champ de la recherche appliquée sur la forêt, il nous semble utile d'inscrire cette

votée en commission qui inclut la mention de l'adaptation des forêts au changement climatique et leur résilience face aux risques.

Ces solutions permettent de bénéficier d'un gain net sur la résilience des forêts et de réduire le risque d'incendie, tout en apportant un bénéfice à la biodiversité locale.

s'agir de la diversification des essences, de la plantation de forêts mélangées, en évitant les monocultures dans les plantations à vocation principale de production de bois, et d'actions de restauration.

La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des bois et forêts, à leur adaptation au changement climatique et aux risques associés, à la promotion de pratiques et itinéraires sylvicoles qui augmentent leur résilience face à ces perturbations,

et ce depuis longtemps- fort heureusement. L'amendement est donc inutile. L'inclusion de ces termes dans l'article pourrait au contraire occulter des solutions locales autres, qui seraient plus pertinentes. J'en profite pour confirmer qu'afin d'accroître l'effort de recherche le Gouvernement a validé un programme exceptionnel de recherche de 50 millions d'euros, qui sera déployé au bénéfice des écosystèmes forestiers, notamment pour leur adaptation au changement climatique. Je mets aux voix

Cet inventaire devrait faire l'objet d'un suivi permanent et être révisé tous les deux ans au minimum. Il serait intégré dans les plans de gestion de la ressource en eau réalisés à l'échelle des bassins versants ou des nappes phréatiques et dans les documents d'urbanisme, permettant ainsi de faciliter la mise en oeuvre des

Il importe d'avoir une cartographie claire de la ressource en eau tenant compte de tous ses usages- eau potable, assainissement, industrie, irrigation, usage récréatif, etc. La notion d'évaluation doit devenir centrale dans la défense incendie. Nous pensons que l'État lui-même doit mener un audit national, département par département, en concertation étroite avec les élus. Cette cartographie serait complémentaire avec la disposition adoptée en commission, qui vise à ce que les besoins de la sécurité civile, en particulier ceux qui concernent la défense des forêts contre les incendies, soient intégrés dans la politique de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

consacré à la Deci, que l'on a évoqué tout à l'heure. Ils sont toutefois largement satisfaits par la proposition de loi issue de ce rapport, qui a été adoptée par le Sénat très récemment.

à la Deci, issue du décret n° 2015-235 du 27 février 2015. Cet objectif, qui ne figure pas dans les dispositions législatives relatives à la Deci, est détaillé dans l'actuelle réglementation à plusieurs reprises.

que des dispositions juridiques de portée nationale interfèrent en la matière. Nous avons confiance en l'intelligence territoriale pour organiser la défense extérieure contre l'incendie dans son ensemble. C'est l'esprit des réformes de la défense extérieure contre l'incendie de 2011 et de 2015. En résumé, sur le plan juridique, cette disposition,

concernés une communication spécifique de leurs obligations. Ensuite, pour aller plus loin que la simple attestation de conformité prévue à l'article 11, nous vous proposons de créer le Dold, le diagnostic de l'obligation légale de débroussaillement. Il s'agit d'un document clair rappelant les informations relatives à la situation des terrains, la la nature des obligations qui incombent à leurs propriétaires et les mesures qu'ils ont prises pour y répondre. Un tel document permettrait à l'ensemble des acteurs d'avoir la preuve de la réalisation des OLD, notamment en cas de mutation d'un terrain.

Nous souhaitons également engager une réflexion sur l'utilisation d'un outil cartographique. Enfin, dans un souci d'efficience, nous proposons de donner la possibilité aux maires, s'ils le souhaitent, d'organiser la mutualisation des OLD des particuliers.

La proposition de loi mentionne, à juste titre, plusieurs outils cartographiques. Leur cohérence est un enjeu majeur, à la fois d'efficacité pour les décideurs et de lisibilité pour les citoyens. Il importe que toutes les mesures prises pour prévenir les feux soient en lien avec l'estimation du risque. La parole est à Mme

plus visibles les périmètres concernés et pour mieux informer les particuliers de l'existence de cette obligation au moment de la délivrance du permis de construire. Cette mesure participera de la pédagogie sur les OLD, ce qui est une bonne chose vu la complexité d'exécution de cette obligation. comme le rappelle l'Assemblée des départements de France, si plusieurs outils cartographiques sont nécessaires, leur cohérence reste un enjeu majeur, à la fois d'efficacité pour les décideurs et de lisibilité pour les citoyens. C'est pourquoi nous proposons, dans un souci de cohérence entre toutes ces procédures et démarches visant à prendre en compte le risque incendie, d'associer les Sdis à la réalisation des documents ou graphiques qui seront annexés aux documents d'urbanisme pour mettre en exergue les OLD. Dans le même ordre d'idée, il nous semble indispensable que cette cartographie soit en cohérence avec la carte d'aléas prévue à l'article 13 du présent texte. Il importe que toutes les mesures prises pour prévenir les feux soient en lien avec l'estimation du risque.

et de maintien en l'état débroussaillé, qui seront annexés aux documents d'urbanisme en application de l'article 8 de la proposition de loi, ne feront que traduire les obligations inscrites dans la loi ou les arrêtés préfectoraux.

qui doivent bien souvent se concentrer davantage sur la protection des habitations que sur la lutte contre le feu. Nous estimons qu'une véritable pédagogie doit être mise en place pour que la prise de conscience soit collective. Chaque particulier doit avoir connaissance de la législation, et donc de ses obligations, mais il doit également comprendre l'intérêt des OLD pour la limitation des départs

ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. Cet amendement vise à compléter ce dispositif par une communication spécifique auprès des propriétaires de terrains concernés.

le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé le terrain concerné, de nombreux citoyens ignorent qu'ils sont soumis à de telles obligations. C'est pourquoi, dans l'esprit de votre amendement, le Gouvernement est favorable à